les réserves d'usage. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie hier sont consultables sur le site du Sénat. Elles seront considérées comme adoptées en l'absence d'observations d'ici à la fin de la séance.- Questions d'actualité

Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat, sur le site internet du Sénat et sur Facebook. Au nom du bureau du Sénat, j'appelle chacun de vous, mes chers collègues, à observer au cours de nos échanges l'une des valeurs essentielles du Sénat : le respect, qu'il s'agisse du respect des uns et des autres ou de celui du temps de parole. La parole est à M. Fabien Gay, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. citoyen et écologiste. Monsieur le Premier ministre, plus d'un million de personnes soutiennent un référendum sur le projet de privatisation d'Aéroports de Paris. Après le scandale des autoroutes et avant celui des barrages hydroélectriques, les Français restent opposés majoritairement au bradage de leur patrimoine commun. Ainsi, 248 parlementaires de tous bords- c'est inédit -se sont associés pour déclencher la procédure du Plus d'un million de personnes soutiennent cette initiative, malgré un site internet complexe, digne du Minitel, malgré une information officielle inexistante, malgré un black-out médiatique assourdissant, sans comparaison avec les millions d'euros d'argent public déboursés pour privatiser la Française des jeux ou organiser le grand débat, et malgré le mépris affiché par le Président de la République, qui n'a pas daigné recevoir les parlementaires signataires. Pourtant, ce soutien apporté par plus d'un million de personnes est une grande victoire démocratique. Le Président de la République, à l'issue du grand débat national, avait promis d'abaisser le seuil du RIP à un million de soutiens. Nous y sommes ! Monsieur le Premier ministre, vous aviez promis de ne pas toucher à la retraite à 62 ans et vous êtes en train de faire passer au forceps une loi qui va faire travailler les Français au minimum jusqu'à 65 ans. Et là, nous sommes un million de soutiens, et vous envisagez de ne pas organiser le référendum Pour redonner confiance en la politique, il est important de tenir ses engagements. Car, si la Constitution ne vous y oblige pas, l'engagement présidentiel vous y invite. Aussi, plutôt que d'utiliser le 49-3 pour étouffer la colère sociale et bâillonner l'opposition parlementaire sur les retraites, êtes-vous prêt à proposer au Président de la République d'utiliser l'article 11, alinéa 1 de la Constitution, pour donner la parole au peuple français sur la privatisation d'Aéroports de Paris ?

j'entends votre question et les remarques qui l'accompagnent, et je ne vous cache pas que je suis un peu surpris par votre lecture du droit actuel.

travers des éléments que vous avez portés à la connaissance du Sénat et qui accompagnent la question que vous posez au Gouvernement, vous faites une lecture que je crois inexacte de la loi constitutionnelle. En premier lieu, il ne vous a pas échappé que la procédure dite « du RIP » exige, pour être mise en oeuvre- je parle

et précis, d'indiquer que l'engagement que nous avons pris de ne pas modifier l'âge légal sera tenu. Je le dis d'autant plus volontiers que les réformes précédentes ont déjà eu pour objet de faire cotiser les Françaises et les Français plus longtemps

peut-être plus discrète, mais pas forcément beaucoup plus respectable, à mon sens. Monsieur le sénateur, il y a un débat parlementaire à l'Assemblée nationale et, demain, il y aura un débat parlementaire au Sénat sur la retraite. Tant mieux ! J'ai eu l'occasion d'indiquer que, dans ce cadre, je ferai usage de l'ensemble des prérogatives qu'offre à un chef de gouvernement la Constitution, comme je suis certain, monsieur le sénateur,

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, jeudi dernier, le ministre de l'agriculture nous annonçait ici qu'un accord européen avait été obtenu pour un budget de la politique agricole commune (PAC), maintenu à 375 milliards d'euros. Il nous disait même que son objectif était désormais d'obtenir 380 milliards d'euros ... En fait, aucun accord n'a été trouvé, et les négociations ont été suspendues. Bref, tout reste à faire Deux questions politiques essentielles demeurent sans réponse. Tout d'abord, quel est l'objectif du Président de la République pour la part française de la PAC ? Depuis 2014, celle-ci est de 9 milliards d'euros par an. Cette somme doit être l'ambition minimale de la France pour ses agriculteurs et les territoires ruraux. Ensuite, quelle PAC voulez-vous ? Le principe de subsidiarité pourrait accroître les distorsions de normes de production entre les États membres, tout en détruisant ce qui reste de commun à notre politique agricole européenne. Quelles orientations entendez-vous donner au plan stratégique national de la France que vous allez soumettre à la Commission ? Sur le verdissement, quelles seront vos priorités ? Et comment allez-vous les articuler avec le de la présidente de la Commission européenne ? Envisagez-vous un renforcement de la conditionnalité des aides ? Souhaitez-vous développer des outils novateurs, comme les paiements pour services environnementaux rendus par les agriculteurs à la société dans son ensemble ? Monsieur le ministre, sur ces questions qui conditionnent son avenir, le monde agricole attend des réponses claires.

Nous nous battons effectivement pour que l'enveloppe française de la PAC ne baisse pas et pour que nos agriculteurs ne soient pas ceux qui financent le Brexit. Le plus fort gage de confiance que l'on peut leur donner, c'est que nous nous refuserons à donner notre accord à tout budget européen qui ferait baisser l'enveloppe dont nous disposons. Nous ne pouvons pas demander plus à nos paysans et leur donner moins de moyens ! Nous n'accepterons jamais une baisse de revenus pour nos agriculteurs : c'est l'engagement du Président ; c'est celui du Gouvernement. La PAC, ce n'est pas trop cher, ce n'est pas, c'est essentiel pour le projet européen que nous voulons, un projet de puissance, un projet de souveraineté alimentaire, un projet de transition écologique. Nous sommes donc fiers, et je crois que nous devons le rester, de produire en Europe des produits de qualité. C'est une mission extrêmement extrêmement importante, et nous devons donner aux agriculteurs les moyens d'y parvenir. Trois points sont encore en discussion, sur lesquels Didier Guillaume mène la négociation. Premièrement, il s'agit de la régulation des marchés, plus que jamais actuelle face aux États-Unis, après le Brexit. Nous devons conserver l'équilibre que propose la Commission entre ceux qui veulent moins de régulations et ceux qui en veulent davantage. Deuxièmement, il s'agit du verdissement, c'est-à-dire de l'architecture environnementale.

de leurs exploitations, car il n'y aura pas de transition si celle-ci n'est pas économiquement viable ; enfin, que soit simplifié le modèle de mise en oeuvre, car, s'il est trop compliqué, les agriculteurs ne peuvent pas s'engager.

La retraite à 85 % du SMIC pour les anciens, que vous avez rejetée ici par un vote bloqué, les suicides, les transmissions et le renouvellement des générations, la régulation du foncier, les zones non traitées (ZNT), qui restent un problème pour tout le monde, la ressource en eau,

Les discussions lors du sommet extraordinaire européen consacré à la négociation du cadre financier pluriannuel ont montré, une fois encore, la complexité de la tâche. L'Union européenne va vraisemblablement devoir gérer de front les négociations avec le Royaume-Uni et celles du budget européen pour la période 2021-2027. La concomitance de ces situations entraîne des risques pour le financement des programmes. Je pense particulièrement au financement de la PAC,

Les sénateurs de l'Aveyron que nous sommes, Jean-Claude Luche et moi-même, ne peuvent que vous transmettre les craintes de nos agriculteurs et de nos concitoyens, bien conscients des enjeux des prochains mois. La baisse de 13 % du budget de la PAC, avec une répartition insatisfaisante entre les deux piliers dans la proposition que le président du Conseil européen avait mise sur la table le 14 février dernier, n'était pas acceptable pour nos territoires. Et je sais que vous partagez ce point de vue.

L'espoir, quant à lui, semble se diriger désormais vers une contre-proposition comme réponse à la crise. La PAC ne peut définitivement pas être une mesure d'ajustement. Chateaubriand disait : « La vieille Europe, elle ne revivra jamais ; la jeune Europe offre-t-elle plus de chances ? » Cette phrase trouve un nouvel écho aujourd'hui. Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous nous détailler les options qui s'offrent à nous, afin de financer ambitieusement la nouvelle PAC, de permettre à l'Union européenne d'offrir, demain, toutes les chances possibles à nos agriculteurs et de défendre notre alimentation ? Car avoir une PAC forte, c'est avoir une Europe forte.

Il faut tirer des leçons de ce Conseil, il faut profondément changer de méthode, il faut repenser notre méthode de travail. Nous ne pouvons pas, au sein de l'Union, décider de crise en crise et laisser des blocs s'affronter. Notre puissance, notre force, c'est notre union, et quand nous organisons la division ou la laissons s'organiser, c'est l'impuissance qui gagne. Nous avons trois priorités avec ce budget européen. Tout d'abord, la politique agricole commune. Je l'ai dit, nous ne pouvons pas demander à nos agriculteurs de faire plus avec moins de moyens. Ensuite, nous voulons de nouveaux instruments de souveraineté, comme le Fonds européen de la défense. Enfin, nous voulons réformer le financement, parce que la solution, ce n'est pas de sacrifier l'agriculteur français pour faire plaisir au contribuable néerlandais, ou de sacrifier l'élu local d'outre-mer pour financer la défense européenne. Cela n'a pas de sens Nous devons, en revanche, augmenter nos ressources et trouver de nouveaux leviers de financement, pour que nous puissions investir en complément des contributions nationales. Si nous disposons des mêmes moyens qu'il y a vingt ans, nous aurons les mêmes politiques qu'il y a vingt ans. Or nous avons de nouvelles ambitions, qu'il faut financer. Comment faire ?

de carbone, le plastique non recyclé, les géants du numérique. Chiche ! Ces taxes sont cohérentes avec nos objectifs politiques, avec l'écologie, avec la justice sociale, avec la protection des Européens. Ce sont de nouvelles ressources, ce sont des armes politiques pour l'Europe.

Les Républicains. Ma question s'adresse au ministre de l'agriculture. Nous avons remis un rapport d'information sur la loi Égalim, adopté à l'unanimité le 30 octobre 2019.

du lait, du boeuf, du porc, des céréales et de la bière, pour ne citer qu'eux. Tous m'ont dit qu'ils souhaitaient voir cette expérimentation prolongée,

que les ambiances dans les box avaient évolué fort favorablement et qu'il se passait quelque chose dans leur filière. Tous reconnaissent aussi qu'il faut aller plus loin,

L'expérimentation prévue dans la loi Égalim se termine le 31 décembre. Il nous faut donc du temps- c'est ce que prévoit le projet de loi ASAP -, pour ajuster cette expérimentation. Nous aurons d'ailleurs le

Union Centriste. Ma question s'adresse à M. le ministre des solidarités et de la santé. Monsieur le ministre, l'inquiétude de nos compatriotes grandit d'heure en heure à mesure que le risque d'une épidémie mondiale se fait jour. jour. Élu de la Haute-Savoie, département touché désormais à plusieurs reprises par des cas de coronavirus, mais aussi frontalier de l'Italie, j'ai été le témoin de la force de notre système de santé, notamment de l'hôpital public. Nous vous soutenons, unanimement je crois, quand, face à cette propagation, vous annoncez le déploiement d'un plan d'urgence national. Si notre économie et notre industrie sont déjà touchées, le spectre du coronavirus dévoile également un autre aspect, tout aussi important à mes yeux, à savoir la fragilité et l'interdépendance de notre économie mondiale, ... Très bien ! ... au centre de laquelle se trouve désormais la Chine. En effet, l'industrie pharmaceutique est fortement affectée par la délocalisation d'une grande partie de sa chaîne de production. Selon l'Académie nationale de pharmacie, quelque 80 % des principes actifs pharmaceutiques utilisés en Europe sont fabriqués hors de l'espace économique européen, et pour une grande partie en Asie.

l'agence nous assure qu'il n'y a aucun problème de pénurie ou d'accès à des médicaments essentiels, que ce soit dans la lutte contre le coronavirus ou pour la prise en charge de maladies aiguës ou chroniques. Cela

depuis plus d'un mois, près de soixante-dix personnes venues de Syrie ou de Palestine se sont installées, dans le dénuement le plus total, sur la place Auguste-Horth à Cayenne. En cours de procédure, les familles syriennes qui bénéficieront, selon toute vraisemblance, du statut de réfugié, subissent directement les conditions d'accueil réservées aux demandeurs d'asile en Guyane. Pour rappel, aucun centre d'accueil des demandeurs d'asile n'est présent sur ce territoire, où l'on a enregistré 3 000 demandes en 2019 et 5 000 Rapportés à la population, ces chiffres font de Cayenne le premier guichet du pays, loin devant l'Île-de-France. En réponse, la loi Asile et immigration a prévu une procédure expérimentale censée réduire l'attractivité de la Guyane. Parallèlement, l'accueil devait être amélioré par la création d'un centre d'hébergement d'urgence, mais l'installation ayant été récemment détruite, tout est à refaire. Vous conviendrez que la situation actuelle ne fait pas honneur à la longue tradition d'asile de la France. Si la procédure adaptée permet de traiter plus efficacement les demandes illégitimes, elle ne doit en aucun cas altérer l'exercice du droit d'asile des personnes nécessitant une protection. Outre les Syriens, je pense aux demandeurs palestiniens, qui voient actuellement leurs demandes rejetées. que nous le voulions ou non, ces populations persécutées continueront d'arriver en Guyane. Encore faut-il que nous soyons capables de les accueillir. Au moment où je vous parle, le centre d'accueil provisoire est déjà saturé, et l'installation prolongée des familles en pleine rue commence à susciter une vive incompréhension. Il nous faut impérativement repenser l'accueil de jour et de nuit et trouver des solutions permettant de désengorger la ville de Cayenne. Monsieur le ministre, quels engagements entendez-vous prendre pour garantir le droit d'asile en Guyane ?

Lors de son déplacement au salon de l'agriculture, le Président de la République, interpellé sur le sujet de la revalorisation des retraites agricoles actuelles, a déclaré : « Tous ceux qui rentreront dans le nouveau système, contrairement à l'ancien, auront une garantie de retraite minimum. Est-ce que je peux vous dire que tous retraités d'aujourd'hui peuvent rentrer ? C'est impossible. C'est impossible, parce que c'est [un coût de] 1,1 milliard d'euros. » Monsieur le ministre, je vous rappelle que, en mai 2018, sur proposition du groupe CRCE, nous avions déjà évoqué le sujet dans cet hémicycle. Alors que le texte présenté, qui proposait de porter le niveau minimal de retraite des exploitants agricoles à 85 % du SMIC, faisait l'objet d'un consensus entre l'Assemblée nationale et le Sénat, l'utilisation du vote bloqué l'avait renvoyé sur la touche. À l'époque, votre gouvernement avait en partie justifié ce choix par la perspective du grand projet de réforme des retraites. Aujourd'hui, nous y sommes. C'est une question de justice et d'équité. Monsieur le ministre, qu'allez-vous faire pour les retraités d'hier et pour tous ceux qui partent dès aujourd'hui ? Avez-vous pensé à la situation des conjoints et des aides familiaux, auxquels leurs pensions permettent à peine de survivre ? Parce que ces agriculteurs, hommes et femmes, ont contribué à faire de notre pays une grande nation agricole, nous leur devons, vous le savez, monsieur le ministre, une solidarité qui soit à la hauteur de leur investissement dans nos campagnes.

Les retraités agricoles touchent des pensions de misère qui découlent de leurs revenus de misère : 780 euros pour les hommes, 590 euros pour les femmes. C'est indécent

Or notre agriculture, c'est une alimentation de qualité, c'est une économie, c'est l'aménagement du territoire, c'est la participation à la transition écologique. Nous devons bien cela à

avant d'être ministre, il a été sénateur. Dans cet hémicycle, nous étions tous favorables à la revalorisation des retraites agricoles, et ce dès 2018, contrairement à votre gouvernement. Nous nous en souvenons bien, puisque Mme Agnès Buzyn nous avait répondu que ce point serait finalement intégré à la réforme des retraites et que vous aviez eu recours au vote bloqué. C'était une façon de dire à la représentation nationale Circulez, il n'y a rien à voir. » Exactement ! Aujourd'hui, à écouter le Président de la République, ce projet de réforme serait révolutionnaire. Il n'en est rien Ceux qui atteindront les 1 000 euros de retraite ne représentent qu'un quart des retraités. Cette retraite minimum ne concernera en réalité que ceux qui ont cotisé

ne concerne finalement que les futurs retraités. Quand allez-vous mettre fin à ce cynisme et à ces effets d'annonce ? Les retraités agricoles touchent les pensions les plus faibles du pays. La retraite moyenne d'un chef d'exploitation après une carrière complète est de 740 euros par mois- 550 euros pour une femme.

quand allez-vous revaloriser les retraites agricoles ? La

transmettra un certain nombre de propositions au Gouvernement, avant l'adoption définitive du texte et/ou du budget de la sécurité sociale que vous aurez à examiner à l'automne prochain. Ces propositions, nous l'espérons, permettront

socialiste et républicain. Ma question s'adresse à M. le ministre des solidarités et de la santé. Monsieur le ministre, on décompte à ce jour plus de 80 000 cas de coronavirus sur la planète et environ 3 000 décès. Chaque jour, de nouveaux lieux, parfois des villes entières, sont confinés. L'épidémie s'étend et commence à toucher notre pays. Pour notre population, ces nouvelles sont évidemment anxiogènes. Elles occasionnent d'ailleurs de déplorables réactions de racisme, que nous condamnons fermement. Nous devons aborder cette épidémie dans un esprit de responsabilité, soucieux de protéger nos concitoyens. Il ne nous faut ni minimiser le risque ni confondre la réalité sanitaire du virus, qui est loin de la grippe espagnole, avec ses effets psychologiques. Cette réalité appelle du sang-froid, sans dramatisation. C'est dans cet esprit que nous souhaitons que le Gouvernement nous apporte des précisions sur la préparation des hôpitaux sélectionnés pour répondre en première ligne. Quels moyens concrets leur sont-ils alloués, à l'heure où la situation de beaucoup d'entre eux est périlleuse en matière de moyens humains et financiers, alors qu'ils sont déjà parfois en grande difficulté pour assumer leurs tâches quotidiennes ? À Paris, les trois hôpitaux désignés sont déjà débordés et ont demandé l'aide des autres établissements hospitaliers. Comment les soignants de ville sont-ils associés aux actions de détection et de suivi des cas ? Vont-ils recevoir des kits de protection ? Enfin, je salue la lettre adressée par le Premier ministre aux maires, bien plus digne et à la hauteur de l'enjeu que la lamentable polémique lancée par l'ex-ministre de la santé sur le sujet. Oui, les élus locaux se retrouvent eux aussi en première ligne. Aussi, qu'attendez-vous concrètement des maires

comme tousser dans sa manche et se laver les mains régulièrement, et il y a des gestes qui peuvent être dévastateurs : les gestes de division, les gestes de repli. C'est pourquoi j'étais hier à Rome, avec mes homologues ministres de la santé européens, pour dire à l'Italie que la France la soutient dans cette épreuve et que nous voulons travailler de façon intelligente, entre partenaires européens, pour trouver des solutions concertées. Nous avons évidemment, à cette occasion, acté qu'il était hors de question de fermer nos frontières. Vous m'interrogez à la fois à la fois sur l'intervention des maires et sur les établissements de santé. S'agissant des maires, vous avez salué la lettre du Premier ministre, et je vous en remercie. Je crois qu'elle était nécessaire. J'ai moi-même eu régulièrement au téléphone, et encore aujourd'hui, de nombreux maires, inquiets lorsqu'il y a une alerte sur leur territoire, ainsi que des présidents d'exécutifs territoriaux, de départements ou de régions. Je continuerai à leur parler, car le rôle des élus, par leur esprit de

plusieurs responsables de syndicats médicaux, hier et encore aujourd'hui, pour les informer que tout le matériel nécessaire leur serait fourni dans les meilleures conditions, au travers du réseau des officines de ville. Une lettre en en voie de finalisation réactualise les consignes et les conseils apportés à l'ensemble des soignants de ville sur le territoire, pour leur dire que faire face à des patients ou à des cas contacts. Quant aux hôpitaux, j'ai souhaité que nous multipliions par trois le nombre d'établissements de santé capables d'accueillir des malades et de les prendre en charge de A à Z, de sorte qu'il n'y a plus aujourd'hui dans notre pays un seul département sans établissement de santé en mesure de prendre en charge ces malades dans de bonnes conditions sanitaires, avec capacité d'isolement, de dépistage, de diagnostic, et avec formation du personnel soignant, médical et paramédical. Je crois que c'est essentiel dans cette période.

votre gouvernement vient de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim, et vous aurez ainsi tenu la promesse de François Hollande faite aux plus radicaux des écologistes. Cette fermeture est un gâchis écologique, économique et humain.

-, un groupe de travail sera créé. La belle affaire ! Tout aurait pu être anticipé ; rien ne l'a été ! Ce territoire est sacrifié. Au-delà du territoire, cette décision dessert les intérêts de notre pays. Tout d'abord, c'est l'argent du contribuable qui va servir à indemniser EDF, à hauteur de 400 millions d'euros. Ensuite, il faudra bien compenser cette perte de production d'électricité. Ainsi, nous devrons allégrement importer plusieurs millions de tonnes de fioul et de gaz, ce qui provoquera un déficit commercial de 2 milliards d'euros par an. Dois-je vous rappeler que l'électricité d'origine nucléaire est en moyenne 80 fois moins productrice de CO2 que celle du charbon, et 40 fois moins que celle du gaz ? Ainsi, la fermeture de Fessenheim se traduira par l'émission de 10 millions de tonnes de CO2 supplémentaires par an. Que faites-vous de tous les discours sur la lutte contre le réchauffement climatique qui ont été tenus Vous me répondrez « éolien ou solaire », mais il faudrait multiplier par quatre les champs éoliens et solaires pour atteindre la cible affichée en 2035 par le Gouvernement. Or Mme Borne a dénoncé, le 18 février dernier au Sénat, un développement anarchique des éoliennes en France Vous pourriez aussi me répondre « biométhane », mais, là encore, les objectifs sont très loin des enjeux réels. Le nucléaire français présente un avantage compétitif sur le plan économique et sur le plan environnemental. ma chère collègue. Pensez-vous que la situation de notre pays et de nos concitoyens soit si florissante que l'on puisse priver la France de ces avantages ?

la fermeture de Fessenheim incarne l'écologie de responsabilité, ... C'est faux ! ... portée par le Président de la République, le Gouvernement et la majorité depuis le début du quinquennat.

la transformation de notre modèle énergétique, vous le savez, en votant la loi Énergie-climat, le Parlement a décidé de ramener le nucléaire à 50 dans notre mix énergétique en 2035. Cela nous conduira évidemment non pas à développer des énergies carbonées, mais à atteindre nos objectifs en matière d'énergies renouvelables. Je voudrais à cet égard souligner que la production d'énergies renouvelables a augmenté de 20 % entre 2018 et 2019. Conformément à la programmation pluriannuelle de l'énergie, les consultations viennent de se terminer, oui, nous allons continuer à augmenter la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique. Dans le même temps, nous accompagnons les territoires, et particulièrement le territoire de Fessenheim, dans cette transformation. C'est le sens du contrat de territoire, qui avait été signé par mon prédécesseur en février dernier. C'est vide ! Comme vous le savez, j'étais sur place avec Emmanuelle Wargon vendredi dernier, et nous avons pu annoncer de nouveaux outils au service du territoire. Nous

Le contraste entre la situation de la France et celle de nos partenaires de la zone euro y est jugé « saisissant ». Hors les effets naturels de la conjoncture, l'État ne fournit aucun effort sur le déficit structurel. C'est pourtant aujourd'hui et maintenant qu'il faudrait agir, compte tenu des taux d'intérêt très bas. Alors que nous nous préparons à examiner le projet de loi portant réforme des retraites, nombre de paramètres financiers demeurent inconnus. Les facteurs d'incertitude se multiplient : intégration des primes des fonctionnaires, revalorisation salariale des enseignants, baisse de la CSG pour les professions libérales et les indépendants. Comment évaluer l'impact budgétaire de ces mesures annoncées au fil de l'eau ? Le financement de la réforme des retraites doit encore être rapproché de celui de la dépendance. Comment arbitrer en effet le niveau des pensions de retraite sans connaître corrélativement l'estimation du coût de la dépendance de nos aînés, ni son impact sur la trajectoire de notre dette publique ? Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner quelques indications sur l'équation budgétaire retenue par le Gouvernement, afin de préserver notre crédibilité en matière de finances publiques ? La

du rapport. Permettez-moi de dire que je ne suis pas d'accord avec votre présentation. La Cour relève bien que nous sommes à 2,2 % de déficit, alors que, lorsque nous avons pris les responsabilités du pays, nous étions à 3,4 % : 0,1 point

avec Olivier Dussopt dans mon ministère. Évidemment, ces efforts paient, et nous avons réduit le déficit. Nous avons aussi été le premier gouvernement à sortir de la procédure de déficit excessif. Certes, la dette reste à un niveau important, et même trop important, comme le ministre de l'économie l'a encore dit très récemment, malgré des taux d'intérêt très bas. En revanche, nous avons « sincérisé » cette dette, ce qu'aucun gouvernement n'avait jusqu'à présent. Vous auriez pu souligner, madame la sénatrice, que la Cour des comptes elle-même révèle que 35 milliards de dettes ont été ajoutés au stock de dettes de notre pays, parce que nous avons fait l'effort, sans précédent, de la réforme

Monsieur le ministre, cela ne peut pas suffire. Vous en conviendrez, le calendrier soutenu des réformes auquel est soumis le Parlement témoigne de votre niveau d'exigence inédit. Cependant, cette exigence doit pouvoir s'exercer dans les deux sens. Aussi, il faut nous accorder les prévisions et les estimations que nous demandons,

organisé par l'association Imagine for Margo et consacré au cancer de l'enfant. Ce fut une journée dense et porteuse d'espoir, car les choses bougent en matière

Après que l'Agence européenne des médicaments a donné l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament innovant, il y a une procédure d'évaluation par la Haute Autorité de santé. Or cette procédure n'est plus adaptée aux médicaments innovants, notamment ceux qui sont destinés aux enfants, en matière, par exemple, de thérapie génique ou de médecine de précision. Une réforme de l'évaluation avait été annoncée. Nous-mêmes, lors de la discussion du dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous avions déposé,

que sont parties toutes les propositions concernant l'accessibilité aux médicaments innovants, y compris sur ce que l'on appelle « l'accès compassionnel » à des thérapeutiques tellement innovantes qu'elles n'ont pas pu être encore évaluées

gagner du temps, des mois, des années de vie, voire pour guérir. Nous vivons une période particulièrement bouleversante à cet égard, car l'accès aux thérapies géniques, grâce aux travaux du Généthon et à la solidarité des Français à travers le Téléthon,

de la formulation qui pourrait être retenue par le Gouvernement dans le cadre, je l'espère, du prochain budget de la sécurité sociale. Je vous tends la main pour que nous puissions mener un travail consensuel sur ces questions, qui dépassent largement les clivages habituels.

Le désarroi des patients, mais aussi des soignants, est grandissant. Nos hôpitaux restent surchargés, nos soignants sont extenués et le manque de lits commence à se faire sentir. Mme Agnès Buzyn, votre prédécesseur, a proposé le plan Ma santé 2022, avec la fin du, la création de 4 000 postes d'assistants médicaux ou, plus récemment, le plan d'urgence annonçant une reprise à hauteur de 10 milliards d'euros de la dette des hôpitaux et un financement supplémentaire de 1,5 milliard d'euros sur trois ans pour l'investissement.

Sont avancées deux hypothèses : soit une approche nationale, soit une reprise régionalisée et, dès lors, un retour par l'intermédiaire des groupements hospitaliers de territoire. Aussi ma question est-elle simple, monsieur le ministre : pouvez-vous nous éclairer sur les modalités et le calendrier de reprise de la dette des hôpitaux

Ma question s'adressait au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, mais le sujet vous concerne aussi, monsieur le ministre des solidarités et de la santé. Vous aurez ainsi une troisième chance de préciser la position du Gouvernement domaine agricole, comme dans la plupart des secteurs, les difficultés pèsent encore plus lourdement sur les femmes. Longtemps rendues invisibles, travaillant sans statut officiel et souvent comme « épouses d'agriculteurs », elles ont obtenu progressivement, mais à force de revendications, des droits sociaux et la mise en place d'un statut de conjoint collaborateur en 1999. Elles représentent aujourd'hui un quart des chefs d'exploitation et des co-exploitants. Si les femmes bénéficient d'une meilleure considération, le chemin reste encore long, surtout en matière de retraite. En 2017, la délégation aux droits des femmes du Sénat a formulé 40 recommandations visant à lutter contre ces difficultés persistantes, notamment en termes d'articulation entre vie professionnelle et familiale et d'accès aux droits sociaux et médicaux fin du travail sans statut, garantie du congé maternité par la mise en place d'un service de remplacement, solutions d'accueil pour la petite enfance en milieu rural et augmentation des retraites. En effet, la moitié des 870 000 femmes retraitées agricoles perçoivent moins de 500 euros par mois en droit propre. Le Gouvernement propose une retraite minimale universelle de 1 000 euros pour une carrière complète au SMIC, mais peu de ces femmes parviennent à se dégager un SMIC, tout au long de leur carrière. Cette mesure ne s'appliquerait en outre qu'aux chefs d'exploitation. En 2018, une proposition de loi portant sur la retraite agricole avançait un minimum de 85 % du SMIC. Elle a été repoussée par le Gouvernement,

de la réforme du régime universel des retraites, cherche justement à améliorer la situation de centaines de milliers de femmes qui se retrouvent en grande difficulté au moment de prendre leur retraite, parce qu'elles ont eu des carrières hachées et sont obligées de travailler jusqu'à 67 ans. Grâce à cette réforme, elles pourront partir plus tôt

la lutte qui se fait chaque jour plus féroce sur les marchés financiers internationaux représente un danger pour nos entreprises françaises. La Banque publique d'investissement, Bpifrance, dont le travail en faveur de l'économie française est à saluer, vient de mettre en place un fonds d'investissement français, dont l'objectif est, justement, de renforcer l'arsenal de notre pays pour protéger ses fleurons face à l'appétit de fonds internationaux aux moyens financiers colossaux. Dénommé « Lac d'argent », ce nouveau fonds d'investissement, dont vous êtes l'instigateur, est un projet louable pour protéger les entreprises françaises. Alors qu'il doit atteindre 10 milliards d'euros, vous ambitionnez de réunir 4 milliards d'euros dès le mois d'avril prochain. Mais voilà que, après avoir constaté que les premiers milliards d'euros ont été levés auprès d'assureurs d'entreprises ou de familles françaises- c'est une bonne chose, je tiens à le dire -, nous apprenons que le fonds Lac d'argent sera alimenté à hauteur de 25 % par un fonds souverain émirati, Mubadala. Même si cet investissement étranger auprès de Bpifrance contribuera au projet de défense de nos fleurons, il soulève certains doutes, que j'aimerais voir éclaircis. Tout d'abord, madame le secrétaire d'État, pouvez-vous nous indiquer quelles garanties vous fixerez concernant, premièrement, la provenance des fonds,

Enfin, ne serait-il pas judicieux d'ouvrir ce fonds d'investissement aux « petits épargnants » français, en toute transparence et par quelque support que ce soit ?

à l'entrée dans le capital, durant toute la gestion de la participation, avec les prises de position qu'elles seront amenées à prendre au moment des assemblées générales, et lors de la cession. Les investisseurs,

La séance est reprise. Je n'ai été saisi d'aucune observation sur les conclusions de la conférence des présidents. Elles sont donc adoptées. J'informe le sénat que des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 L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote sur la deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture, visant à améliorer l'accès à la prestation de compensation du handicap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

Le 3 octobre dernier, vous déposiez, monsieur le président Milon, cette proposition de loi, à l'appui des travaux conduits par le sénateur Philippe Mouiller, avant une adoption en première lecture par votre chambre, à l'unanimité, le 5 novembre. ce texte à l'Assemblée nationale le 15 janvier a ensuite permis d'enrichir celui-ci, en ses articles 2 et 4- j'en profite pour rendre hommage à votre collègue député Philippe Berta, qui s'était déjà par le passé saisi de cette question. de loi à l'unanimité est le signe, je le crois, d'une reconnaissance de sa qualité. Votre commission des affaires sociales a adopté ce texte modifié, là encore, à l'unanimité, ne laissant plus aujourd'hui place qu'aux explications de vote et au vote. En cinq mois donc, nous aurons fait évoluer positivement plusieurs dispositions d'importance relatives à la prestation de compensation du handicap (PCH). Je crois que nous pouvons nous féliciter collectivement de cette célérité et de cet esprit qui nous ont animés. J'ai eu l'occasion de le rappeler la semaine dernière devant un certain nombre d'entre vous, le travail engagé s'est aussi prolongé sur le champ de la compensation du handicap, avec des annonces fortes du Président de la République le 11 février dernier à l'occasion de la Conférence nationale du handicap. Tout d'abord, nous rouvrons pour la première fois le périmètre des besoins compensés par la prestation avec, au 1 janvier 2021, son élargissement aux besoins attachés aux parents en situation de handicap d'enfants jusqu'à 7 ans. C'est un investissement de 184 millions d'euros que nous réalisons pour que le handicap ne soit plus un obstacle au projet parental, qu'il ne soit plus source de renoncement à une vie à laquelle tout un chacun Aussi, il sera bientôt mis fin à la situation ubuesque selon laquelle une personne en situation de handicap peut être accompagnée pour se nourrir, mais, dans le même temps, pas pour laver sa vaisselle. Enfin, nous allons engager un travail pour identifier concrètement les évolutions qui doivent s'attacher à la prestation de compensation du handicap pour une meilleure prise en compte des handicaps psychiques et du trouble du neuro-développement. nous parlions, lors de l'examen de ce texte en commission, de l'importance de la nécessaire coconstruction qui doit animer tant l'État que les collectivités territoriales, au premier rang desquelles l'Assemblée des départements de France Je connais, mesdames, messieurs les sénateurs, votre attachement aux départements ; c'est effectivement ensemble que nous réussirons. L'accord de méthode signé voilà deux semaines entre l'État, l'Assemblée des départements de France, les fédérations et associations gestionnaires de l'offre médico-sociale constitue à ce titre un acte important,

au plus proche des besoins des personnes et garantes de la maîtrise des délais pour l'attribution des droits. Cette exigence, nous devons nous la fixer collectivement, là où nous nous sommes trop habitués aux difficultés. L'État sera exigeant concernant l'équité de traitement sur le territoire, et soutiendra aussi, y compris financièrement, cette ambition. Oui, il reste encore à faire, mais je veux croire que le chemin que nous prenons est le bon, à l'image de la proposition de loi qui nous est présentée aujourd'hui et dont je souhaite rappeler les principes. L'article 1 du texte supprime une barrière d'âge. Cette nouvelle rédaction permet aux personnes en situation de handicap n'ayant pas formulé de demande de prestation de compensation du handicap

et la portée. L'article 2 contribue à l'évolution du dispositif relatif aux fonds de compensation. Il ouvrira la voie à un décret, pris dans les six mois suivant l'adoption de la loi- j'ai réaffirmé ce principe devant votre commission la semaine dernière -, qui fixera l'emploi de ces fonds, en concertation avec les associations. Au-delà de la parole du Gouvernement, l'adoption, lors de la discussion à l'Assemblée nationale, d'un amendement qui tend à proposer au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport dans les dix-huit mois suivant l'application du décret, est un gage de notre volonté commune. L'article 3 vise à inclure la PCH dans le corpus des droits à vie, dès lors que le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement. Il est la continuité de notre objectif de double simplification, à la fois celle- majeure -de la vie des personnes en situation de handicap aux parcours parfois révoltants, mais aussi celle des MDPH, qui pourront se recentrer sur leur mission d'accompagnement et de conseil des personnes en situation de handicap. enfin, à l'article 4, dont la rédaction initiale a été enrichie lors de la première lecture au Sénat pour englober la question des transports, mais aussi, sur l'initiative de la sénatrice Patricia Schillinger, celle de la compensation du handicap pour les enfants.

de la cité inclusive que nous souhaitons, de la pleine intégration des personnes en situation de handicap dans le droit commun autant que faire se peut, sans créer de chemins parallèles entre les personnes en situation de handicap et les les autres. Sur la question des enfants, je souhaite, là aussi, rappeler que nous avons pris des engagements nouveaux lors de la Conférence nationale du handicap, qui constituent des éléments de réponse importants aux difficultés plusieurs fois soulevées, notamment dans le rapport récent de Daniel Lenoir. D'une part, nous étendrons l'année prochaine le forfait d'intervention précoce mis en place au titre de la stratégie nationale pour l'autisme au sein du trouble du neuro-développement à l'ensemble des enfants de 7 à 12 ans. Cela permettra notamment d'apporter une réponse plus rapide et plus structurée aux enfants qui souffrent de troubles dys ou de troubles de l'apprentissage, que nous ne pouvons laisser sans accompagnement. D'autre part, mais c'est un chantier qui va nous prendre un peu de temps, nous souhaitons, d'ici à 2022, être en mesure de proposer un parcours de soins de rééducation à tous les enfants en situation de handicap ou souffrant de suites de maladies lourdes, avec une prise en charge par l'assurance maladie et une exigence de qualité.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, si l'adoption imminente de cette proposition de loi fournit des motifs de satisfaction certains, le contexte de la discussion de ce texte, quant à lui, doit nous pousser à la réflexion. Je commencerai par les motifs de satisfaction, qui sont nombreux. Il faut d'abord se réjouir qu'une initiative parlementaire soit adoptée si rapidement. Déposée au Sénat le 3 octobre dernier, cette proposition de loi a été adoptée à l'unanimité en séance publique le 5 novembre, puis examinée en commission à l'Assemblée nationale le 18 décembre, si bien que les députés ont pu l'adopter en séance plénière, à l'unanimité également, le 15 janvier dernier. Transmis au Sénat, le texte a fait l'objet d'une nouvelle unanimité mercredi dernier, après avoir été examiné selon la procédure de législation en commission. Il faut se réjouir aussi des apports de nos collègues députés et ainsi du bon fonctionnement du bicamérisme, même si l'on peut s'étonner qu'une deuxième lecture ait été rendue nécessaire, alors que nos vues convergeaient manifestement depuis l'origine. Les dispositions contenues dans ce texte sont autant d'avancées significatives pour les personnes handicapées et leurs familles. Je les rappellerai brièvement. L'article 1 supprime la barrière d'âge de 75 ans pour déposer une demande de prestation. Il a été voté conforme par nos collègues députés ; nous n'y reviendrons donc pas. L'article 2 rend opérationnels les fonds départementaux de compensation du handicap en clarifiant leur base légale, ce qui permettra au Gouvernement de prendre le décret d'application tant attendu. Les députés ont ajouté une demande de rapport sur la mise en oeuvre de ce dernier et l'évolution du reste à charge des personnes ayant déposé au moins une demande auprès d'un fonds départemental. C'est, en l'espèce, un moyen d'évaluation sans doute utile, quoi que l'on puisse penser, en général, des demandes de rapport. L'article 3, qui crée un droit à vie à la PCH lorsque c'est possible, simplifie les démarches des bénéficiaires ainsi que le contrôle de l'utilisation de la prestation, a été adopté avec quelques modifications rédactionnelles. L'article 4, enfin, crée un comité stratégique chargé de formuler des propositions pour améliorer la prise en charge des transports des personnes handicapées. Le périmètre de sa réflexion a été élargi, au Sénat puis à l'Assemblée nationale, aux besoins des enfants et à la considération de tous les types de mobilités. À cet article, nous aurions tous souhaité un dispositif plus consistant, mais vous savez bien, chers collègues, à quelles limites constitutionnelles sont confrontés les parlementaires. Par ailleurs, la meilleure preuve de l'utilité d'un tel organe de réflexion et de proposition est donnée par la lecture des engagements récents du Gouvernement à l'issue de la Conférence nationale du handicap, puisque la mobilité n'en fait pas partie ... Je le souligne non pas par malice, mais pour que la probable unanimité sur ce texte ne nous masque pas les efforts qui restent à accomplir. Les conclusions de la Conférence nationale du handicap sont significatives, mais elles ne sauraient être définitives. À certains égards, la question des barrières d'âge se pose à nouveaux frais.

Étant par ailleurs moins souvent en emploi, ces personnes passent en moyenne 8,5 années sans emploi ni retraite après 50 ans, soit près de 7 ans de plus que les personnes sans incapacité, et cet écart s'accroît Cette curieuse situation s'explique par le fait que les personnes sans handicap bénéficient plus aisément de certains dispositifs, du type « carrières longues ». Alors que le Gouvernement nous somme de consentir à échafauder un nouveau système, tâchons de conserver une vision cohérente de la politique destinée aux personnes handicapées, en articulant compensation, prévention et garantie des ressources. Mais à chaque jour suffit sa peine : pour l'instant, soyons fiers, mes chers collègues, de voter cette nouvelle avancée en faveur des personnes handicapées et de leurs familles. Ne perdons cependant pas de vue l'ampleur des défis qui restent à relever, et, surtout, ne doutons jamais des apports indispensables du Parlement à l'amélioration de nos politiques publiques ! La parole est à Mme Cathy

cette proposition de loi déposée par le groupe Les Républicains supprime la barrière d'âge pour la PCH avant laquelle les personnes doivent déposer leur demande de prestation de compensation du handicap reconnu avant l'âge de 60 ans. Jusqu'à présent, les personnes concernées devaient entamer la démarche avant 75 ans, mais depuis des années, les associations de personnes en situation de handicap militent pour supprimer cette barrière qui restreint injustement les droits de celles-ci. En reprenant la proposition de supprimer la limite de 75 ans, ce texte constitue un progrès pour les personnes qui ne seront plus soumises à cette contrainte administrative.

Il y a urgence à améliorer le dispositif de compensation du handicap, en permettant le financement de l'accès aux aides techniques et humaines dont les barèmes n'ont pas bougé depuis quinze De la même manière, le périmètre des prestations doit être élargi comme le demande Arnaud de Broca, président du Collectif Handicaps, puisque, « aujourd'hui, les prestations prennent en compte l'achat d'un fauteuil roulant, mais pas le financement d'aides ménagères L'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap passe également par la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). À grand renfort de communication, le Gouvernement avait annoncé la revalorisation de l'AAH à 900 euros, alors même que ce plafond demeure au-dessous du seuil de pauvreté.

alors que la majorité à l'Assemblée nationale, contre l'avis du Gouvernement, a adopté un texte en ce sens le 13 février. Il s'agit d'un sujet qui préoccupe de nombreux couples, car la relation de dépendance financière et psychologique entre la personne en situation de handicap et sa conjointe ou son conjoint remet en cause l'autonomie de cette personne. Il convient de rappeler que l'AAH n'est pas un minimum social comme un autre : cette allocation a pour objet de venir au secours d'une personne qui, du fait de son invalidité, se trouve dans la stricte impossibilité de disposer de ressources suffisantes liées au travail. Comme elle nous l'a écrit, l'association Cap'devant

Comme en première lecture, le groupe CRCE votera en faveur de cette proposition de loi, qui démontre par ailleurs l'utilité de l'initiative parlementaire, alors même que le Gouvernement remet en question les droits d'expression des groupes parlementaires

afin de mieux couvrir l'ensemble des besoins des bénéficiaires. Notre assemblée se réunit aujourd'hui pour voter la proposition de loi visant à améliorer l'accès à cette prestation. La PCH

de besoins particuliers : aide humaine, aides techniques, aménagement de logements et de voitures, allocation pour l'éducation, entretien, chiens guides, etc. Ce dispositif appelle des améliorations. Il s'agit notamment de simplifier les modalités d'attribution de la prestation, jugées trop complexes, et d'améliorer le contrôle de son utilisation par les départements.

L'article 1 supprime la barrière d'âge fixée à 75 ans. Il s'agit là d'une amélioration importante pour rendre la prestation plus accessible. Le dispositif actuel excluait les personnes qui n'avaient pas jugé opportun de demander cette prestation

L'article 2 améliore l'encadrement des fonds de compensation du handicap gérés par les départements. Il clarifie la base légale de ces fonds, ce qui va permettre de sécuriser le dispositif, de le rendre plus facilement applicable et de diminuer le montant du reste à charge pour les bénéficiaires. L'article 3 pérennise à vie l'attribution de la PCH en cas d'absence d'évolution prévisible du handicap. En outre, il simplifie les durées d'attribution des différents éléments qui composent la prestation en les harmonisant sur une période de dix ans.

Madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, ces dispositions contribueront à améliorer de façon certaine le quotidien des personnes touchées par un handicap.

Le second, plus nuancé, est une forme d'incompréhension. Ce texte aurait pu être inscrit dans le marbre il y a plus d'un mois, et nous votons aujourd'hui une proposition de loi qui, presque à la virgule près, est identique

Nous pouvons nous étonner qu'une demande de rapport soit désormais formulée à l'article 2, sachant que le Sénat se prononce en faveur d'une réduction de telles demandes, en raison de leur visibilité parfois incertaine.

Offrir la possibilité à chaque personne de devenir parent, c'est l'honneur de la France. Nous soutenons ces annonces, car il nous appartient collectivement de relever ces défis car le quotidien des personnes en situation de handicap et de ceux qui les accompagnent n'est pas à prendre à la légère, bien au contraire ; car chaque jour est important pour rendre enfin possible l'impossible.

Aussi, je m'arrêterai brièvement sur deux points. Tout d'abord, l'article 1 témoigne de l'importance de ce texte et répond à un principe de justice sociale en supprimant une limite d'âge dont la justification demeurait difficilement compréhensible pour les bénéficiaires de la PCH.

en remercie. Les durées d'attribution des différents éléments de la prestation, hors aide humaine, sont ainsi homogénéisées. C'est une étape importante, qu'il convient de souligner.

En effet, la couverture des frais de transport par la PCH pose de réels problèmes aux intéressés, notamment lorsque les structures médico-sociales ne sont pas présentes dans leur département de résidence. Cette situation est susceptible de limiter leur accès aux soins ou d'avoir une incidence non négligeable sur leurs liens familiaux, par exemple.

se trouver en situation de handicap, c'est se heurter au quotidien à des obstacles majeurs supplémentaires ; c'est avoir besoin d'aide, d'équipements et d'aménagements. Tout cela représente un coût c'est pour la prise en charge de ces besoins qu'intervient la prestation de compensation du handicap. Cette aide personnalisée versée par les départements constitue l'un des dispositifs importants de la loi du 11 février 2005.

Néanmoins, nous n'ignorons pas la réalité vécue par les personnes en situation de handicap et par leurs familles. Les délais d'instruction des demandes et des décisions relatives à l'attribution de la PCH sont encore beaucoup trop longs et varient grandement d'un département à l'autre. outre, l'on retrouve ces inégalités territoriales dans les critères d'éligibilité des bénéficiaires, très hétérogènes, comme dans les montants versés, trop variables d'un département à l'autre.

la PCH répond insuffisamment aux besoins spécifiques des enfants en situation de handicap et des personnes souffrant d'un handicap psychique. Enfin, les personnes dont le handicap survient après 59 ans ne peuvent prétendre à cette prestation. Il conviendrait de supprimer la barrière des 60 ans : dans les faits, un handicap survenu après cet âge sera traité au titre du vieillissement, donc avec une prise en charge beaucoup moins favorable. me conduisent à évoquer deux sujets liés à l'actualité récente. Ils préoccupent beaucoup les personnes en situation de handicap, leurs familles et leurs représentants.

pour continuer à bénéficier normalement de cette aide. Je ne peux donc que saluer les mesures adoptées, le 13 février dernier, contre l'avis du Gouvernement et de la majorité à l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment de supprimer la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l'AAH et de relever l'âge maximal pour bénéficier de la PCH.

ont claqué la porte de ce qu'elles ont appelé « un simulacre de concertation » organisée par le Gouvernement. Elles considèrent, avec juste raison, que l'AAH n'est pas un minimum social comme les autres : ce sont les conséquences des déficiences et des incapacités qui fondent l'accès à cette allocation et non la situation de vulnérabilité sociale.

Cette fusion de l'AAH dans le RUA, si elle était confirmée, dégraderait les droits des personnes en situation de handicap. Les logiques comptables et de rationalisation des politiques publiques suivies par le Gouvernement vont finir par ériger un modèle de société dans lequel les spécificités du handicap ne sont pas suffisamment prises en compte. Dès lors, la mise à l'écart et l'isolement des personnes seraient encore aggravés. Ce n'est évidemment pas notre vision de ce que doit être une société inclusive, qui s'enrichit des différences et permet à chacun de choisir sa vie.

pour citer un ancien Premier ministre, dont les idées n'étaient pas les miennes, mais dont j'appréciais l'art de la formule, « notre route est droite, mais la pente est forte ». Cette phrase illustre assez bien les enjeux du sujet qui nous réunit aujourd'hui : l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap. si nous avons un cap et une trajectoire- des intentions, en tout cas -, le moins que l'on puisse dire est que le chemin pour les atteindre ressemble plus à l'ascension du mont Ventoux qu'à la circulation tranquille à bicyclette à travers mes chères plaines d'Artois Bien sûr, à l'instar de mes collègues de la commission des affaires sociales, je me félicite que ce texte parvienne à son terme, dans un climat de consensus entre nos diverses sensibilités politiques comme entre nos deux assemblées. Néanmoins, beaucoup trop encore reste à faire, quinze ans après une loi dite « fondatrice », qui devait inscrire dans le marbre la compensation de chaque handicap, apporter une réponse à chacune de ses problématiques et créer une société véritablement accessible et inclusive.

que le chantier annoncé, et je l'espère bientôt ouvert, du projet de loi relatif au grand âge offre l'occasion de remettre en débat la réflexion sur une prestation unique et universelle, destinée à compenser toutes les formes de perte d'autonomie, qu'elles soient dues au vieillissement ou au handicap.

Elles sont les bienvenues, mais, comme certains de mes collègues, je me dois d'alerter quant aux capacités financières dont devront disposer les départements pour garantir l'efficacité de ces fonds.

un meilleur remboursement des coûts des dispositifs médicaux, un programme national pour l'innovation technologique. Mais, vous le savez comme moi, c'est la question de l'engagement financier de l'État qui reste au centre. la mobilisation des acteurs, le changement de regard, la mise en accessibilité, ou encore l'adaptation se feront si les moyens débloqués sont à la hauteur du long chemin qu'il nous reste à parcourir. Les mois qui viennent seront déterminants pour constater la mise en actes de ces intentions, dont je ne doute pas de la sincérité. D'ailleurs, nous aurons nombre d'occasions de les mettre à l'épreuve les conclusions de la mission confiée à Philippe Denormandie sur les aides techniques et de la mission relative au logement inclusif ; les travaux du comité stratégique consacré aux transports ; le sort réservé à la proposition de loi portant suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans la base de calcul

nous examinons aujourd'hui une proposition de loi, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, visant à améliorer l'accès à la prestation de compensation du handicap. Créée par la loi du 11 février 2005, cette prestation bénéficie actuellement à près de 350 000 enfants et adultes en situation de handicap ; elle les aide à faire face aux frais liés à leur situation. Malgré une prise de conscience par les pouvoirs publics des difficultés financières liées au handicap- les dépenses en faveur des personnes en situation de handicap ont progressé de 13,5 milliards d'euros entre 2005 et 2014 -, on constate que de réelles injustices perdurent : il est du devoir du législateur de les faire cesser.

L'adoption de cette proposition de loi à l'unanimité par nos collègues députés démontre, une nouvelle fois, la prise de conscience de la société vis-à-vis du handicap et des difficultés liées à celui-ci.

En supprimant la barrière d'âge pour étendre l'éligibilité à la prestation de compensation du handicap au-delà de 75 ans, il répond à une véritable demande du monde du handicap. en effet, le passage à l'allocation personnalisée d'autonomie peut laisser penser que le handicap cesserait à 75 ans pour faire place à la perte d'autonomie. Or c'est évidemment faux, les deux phénomènes étant nettement dissociables. (IGAS), dans son rapport de novembre 2016 sur l'évolution de la prestation de compensation du handicap, avait souligné que l'évolution des limites d'âge constituait une piste d'amélioration majeure.

résultera un réel gain de temps pour un public vulnérable, grâce à la simplification de démarches administratives parfois très pesantes. Le 11 février dernier, dans le cadre de la Conférence nationale du handicap, le Président de la République a lancé un appel à la mobilisation nationale autour du handicap, prenant un certain nombre d'engagements au service des objectifs énoncés dans cette proposition de loi. Je pense notamment à l'exonération totale de cotisations sociales sur le dédommagement de l'aidant financé sur la PCH, ainsi qu'à la mise en place d'une garantie délai pour l'octroi des prestations. Enfin, nous nous réjouissons que la proposition de loi organise la réflexion préalable à une prise en charge enfin intégrée des transports des personnes handicapées,

la rigidité de sa mise en oeuvre et son inaptitude à couvrir l'ensemble des besoins de la personne. De fait, la permanence de restes à charge élevés, le maintien de barrières d'âge à 60 et 75 ans

un second comité stratégique serait mis en place, destiné à proposer des évolutions des modes de transport des personnes handicapées dans le cadre d'une gestion logistique et financière intégrée.

pour travailler sur toutes les zones frontières et sur l'articulation de l'AAH avec les prestations, notamment relatives au logement.

L'ordre du jour appelle la discussion, en nouvelle lecture, de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, visant à lutter contre les contenus haineux sur internet

Là où le bât blesse, c'est que ce retrait n'est pas mis en oeuvre, ou alors à des conditions à la main des réseaux sociaux, ce dont la puissance publique ne peut se satisfaire. Dans ce contexte, que prévoit la proposition de prompt retrait, notamment par la création d'un délit autonome complété par un dispositif de régulation et de supervision tout à fait inédit, confié au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), qui doit introduire des règles et de la transparence là où règne aujourd'hui la plus grande opacité. Il est temps de demander à ces réseaux sociaux des comptes sur la manière dont ils décident de retirer ou non les contenus mis en ligne par nos concitoyens. Il est temps de leur imposer des exigences à la hauteur du rôle et de l'emprise qui,, sont aujourd'hui les leurs dans nos démocraties, et face auxquels le n'est pas tenable. initiative, je tiens à le souligner, n'a pas encore d'équivalent, puisque, à la différence de la loi adoptée en Allemagne, elle repose sur un véritable dispositif de supervision par une autorité administrative indépendante, destiné à assurer un dialogue étroit avec les acteurs concernés, à décliner de manière opérationnelle la future loi et à en garantir une application efficace. Pour autant, ce texte ne s'en remet pas à la seule régulation des réseaux sociaux pour faire appliquer nos lois. Parallèlement à l'instauration de ces nouvelles règles, c'est notre arsenal judiciaire qui sera progressivement modernisé, avec la mise en place d'un parquet spécialisé dans les infractions commises en ligne et le déploiement progressif de dispositifs de plainte en ligne. Cette mise à niveau est absolument cruciale pour agir efficacement contre l'impunité qui prévaut actuellement en ligne ; le Gouvernement est pleinement mobilisé pour y parvenir. Je ne m'explique pas- ou, peut-être, je me l'explique trop bien -comment une écriture de compromis n'a pu être trouvée entre les deux assemblées, sur un sujet où le consensus était à portée de main

Puisque nous sommes en nouvelle lecture, en sorte que chacun connaît déjà les tenants et aboutissants de la discussion, permettez-moi d'en venir directement à ce qui fait débat entre nous- à tout le moins, entre le Gouvernement et la majorité sénatoriale.

C'est notamment pour cette raison que le texte a largement évolué par rapport à sa première version, après son passage au Conseil d'État et en première lecture à l'Assemblée nationale, mais aussi en première lecture au Sénat, dont nombre des ajouts ont été conservés par les députés en nouvelle lecture.

Ils relèvent, à chaque fois, d'une application rigoureuse des conditions générales d'utilisation des plateformes concernées, non de la loi. Le texte transmis au Sénat en nouvelle lecture est équilibré : il a été adapté et mieux calibré pour répondre aux préoccupations de la Commission européenne tout en restant ambitieux.

J'ajoute que c'est une bien mauvaise bataille, à mes yeux, de lancer l'offensive de manière circonstancielle, à un moment où la classe politique se sentirait menacée. Ce qui doit nous presser, c'est l'affaire Noisiel, l'affaire Mila, l'explosion du cyberharcèlement et de la haine en ligne, pas l'affaire Griveaux,

Pourtant, alors même que, dans d'autres domaines, à mes yeux moins vitaux- au sens propre du terme-, vous ne cessez d'en appeler à des actions audacieuses, à une régulation forte, vous semblez, en la matière, vous satisfaire d'une forme de au lieu de soutenir ce premier pas législatif

Tenir des propos haineux et illicites en ligne ne relève pas de la liberté d'expression ; c'est un délit, qui doit être sanctionné. Il nous faut par ailleurs, me semble-t-il, appréhender le texte que nous examinons aujourd'hui dans un contexte plus large, et en saisir toute la portée. Comment ne pas voir la menace qui plane sur nos institutions démocratiques elles-mêmes ? S'il y a un élément au regard duquel les événements survenus dans le cadre de la campagne de l'élection municipale parisienne doivent collectivement nous interpeller, c'est bien la nécessité que nos outils et nos lois s'adaptent enfin à l'ère du numérique. Bien sûr, ce texte n'aurait rien empêché à l'épisode en question. Mais il est urgent que l'État montre et démontre qu'il est capable de protéger efficacement ses citoyens, en ligne comme hors ligne. Il y a, en la matière, une continuité dans l'action de ce gouvernement je pense notamment à l'introduction de la plainte en ligne, qui sera expérimentée dès cette année, à la spécialisation d'un parquet en matière numérique, qui permettra de mieux combattre les abus en ligne et de gérer plus efficacement les échanges avec les réseaux sociaux, et à la proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui pour enfin lutter contre les contenus haineux sur internet. C'est dans ce même souci d'efficacité que la France se bat pour que soit mis en place à l'échelon européen un véritable cadre de supervision des réseaux sociaux en matière de contenus dangereux. Comme le président Larcher, qui a eu, en l'espèce, des mots justes, je vous propose de mettre un coup d'arrêt à ces « torrents de boue » qui n'ont rien de virtuel et qui, détruisant quotidiennement des réputations et des vies, finissent par salir notre démocratie dans son ensemble. La puissance publique ne doit pas avoir la main qui tremble au moment de prévoir des sanctions sévères à l'encontre des plateformes et des réseaux qui ne se mettront pas à niveau pour protéger nos concitoyens. Ce qui est ici en jeu, en effet, ce n'est pas seulement notre vie en ligne ; c'est le c'est le respect de la dignité des personnes, le respect de l'État, le respect de la loi, le respect de tout ce qui fait tenir notre société. Ce qui est en jeu, c'est le début d'une forme de reconquête républicaine. La parole

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le Sénat est saisi en nouvelle lecture de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet. l'examen de ce texte en première lecture dans un esprit ouvert et constructif ; nous partageons tous, monsieur le secrétaire d'État, l'objectif poursuivi, et de nombreuses améliorations ont été adoptées en commission et en séance grâce aux amendements émanant de la quasi-totalité des groupes politiques de notre assemblée. Examinée, hélas, selon la procédure accélérée, cette proposition de loi n'a fait l'objet que d'une seule lecture par l'Assemblée nationale puis par le Sénat avant la réunion d'une commission mixte paritaire. Nous n'avions pas eu d'étude d'impact ; nous n'avons pas eu non plus de véritable navette navette ! Je l'ai dit et je le redis : je regrette vivement cette précipitation. Elle a desservi le rapprochement des positions et ne semble sérieusement justifiée par aucune contrainte de calendrier. La réflexion sur ce texte a été engagée il y a plus de deux ans,

Malgré un travail constructif entre rapporteurs- je tiens à souligner l'excellence du dialogue que nous avons pu entretenir, Mme Laetitia Avia et moi -, cette commission mixte paritaire a constaté qu'elle ne pouvait élaborer un texte commun. la principale divergence avec les députés restait la rédaction retenue par l'Assemblée nationale pour l'article 1, la création d'un nouveau délit- ce n'est pas une mince affaire ... -, et ce en dépit d'un large consensus sur tout le reste, la régulation des plateformes comme le renforcement de la prévention et des outils judiciaires contenus relevant de la haine en ligne. Preuve d'une large convergence de vues entre les deux chambres, l'Assemblée nationale a conservé de nombreux apports du Sénat lors de la nouvelle lecture. Je m'en réjouis ! La position du Sénat n'a jamais été de bloquer ce texte ou de le « détricoter », mais il s'agissait bien de le renforcer et de le sauver des risques d'inconstitutionnalité Grâce à nous, les modalités générales de notification des contenus illicites aux hébergeurs ont été précisées, afin d'être rendues plus aisées à manier pour les internautes, tout en restant pleinement respectueuses du droit européen. Les principaux apports du Sénat pour sécuriser juridiquement la régulation des grandes plateformes ont aussi été conservés. Nous avons ainsi précisé les nouvelles obligations de moyens, strictement proportionnées à l'objectif de préservation de la dignité humaine, en interdisant toute obligation de surveillance générale des réseaux. Nous avons aussi renforcé les pouvoirs de contrôle- accès aux algorithmes -et de sanction- publicité des décisions,

que de corrections formelles. Enfin, des ajouts introduits au Sénat et destinés à s'attaquer à des sujets laissés de côté par le texte initial ont été conservés ou confortés : lutte contre le financement des sites haineux et lutte contre la viralité, les plateformes étant encouragées à limiter les fonctionnalités de partage et l'exposition du public

du caractère inabouti de leur réflexion, les députés ont modifié, et ce pour la quatrième fois, la définition d'un « contenu haineux ». Ils ont maintenu l'ajout du négationnisme proposé par le Sénat, mais ils ont exclu les infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme ... qu'ils avaient pourtant eux-mêmes introduites en première lecture ! De manière plus surprenante, ils ont exclu l'exposition des mineurs à des messages violents, incitant au terrorisme, ou à des jeux dangereux, tout en conservant l'exposition des mineurs à des messages pornographiques. Où est la cohérence ? Très bien ! La commission des lois a supprimé ce dispositif pénal : probablement contraire au droit européen et déséquilibré au détriment de la liberté d'expression, il incitera immanquablement les plateformes à censurer par prudence des contenus pourtant pourtant licites. Le Sénat n'est pas le seul à alerter sur les inévitables effets pervers de cette disposition. De très nombreux acteurs de la société civile en demandent la suppression : la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le Conseil national du numérique, l'ordre des avocats, le rapporteur spécial de l'ONU, et même l'Inter-LGBT tous nous ont fait part de leurs inquiétudes ! Les entreprises du numérique ne sont pas en reste : non seulement les géants américains, qui sont farouchement contre- on pouvait s'y attendre ! -, mais aussi nos propres champions français du numérique- cela devrait vous alerter, monsieur le secrétaire d'État chargé du numérique ! Hier Hier encore, dans une tribune, le moteur de recherche Qwant exhortait le législateur à renoncer à l'obligation pénale de retrait en vingt-quatre heures, pointant le risque d'inconstitutionnalité ! En Allemagne, en décembre dernier, le ministre fédéral de la justice a annoncé vouloir réviser la loi relative aux réseaux sociaux, loi NetzDG, pour les intimes, pour lutter contre la multiplication des retraits abusifs de contenus pourtant licites ; devons-nous vraiment faire la même erreur ? C'est toute la question posée par cet article 1. Je veux le souligner avec force : le Sénat ne s'est évidemment pas résolu à l'inaction face aux grandes plateformes. Mais nous privilégions les solutions efficaces, et surtout applicables, celles qui conservent toute sa place à la puissance publique, la régulation du CSA, plutôt que des innovations incertaines déléguant toujours plus de pouvoir aux géants américains du numérique. Ce n'est pas à eux d'exercer la police de la liberté d'expression ! La commission des lois a donc réaffirmé que le délai de vingt-quatre heures pour le retrait d'un contenu manifestement haineux devra être un objectif à atteindre pour pour les grandes plateformes, consacrant ainsi une obligation juridique de moyens. Pour s'assurer du respect de cette obligation, le régulateur se voit d'ailleurs confier de solides pouvoirs de contrôle, passant au besoin par la communication des algorithmes utilisés, et de sanction, l'amende administrative pouvant aller jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel. Avec la version du Sénat, les réseaux sociaux devront bien rendre des comptes à leurs utilisateurs et prouver qu'ils consacrent suffisamment de ressources humaines et techniques à la satisfaction de cet objectif. La La commission des lois a en outre rétabli plusieurs dispositions qui, supprimées par l'Assemblée nationale, permettent pourtant de s'attaquer aux ressorts profonds de la diffusion de la haine en ligne.

la mission du CSA consistant à encourager la lutte contre les faux comptes qui, sur les réseaux sociaux, ne sont dédiés qu'à la propagation de contenus haineux illicites, les fameuses « fermes à trolls a été réaffirmée la mission du CSA en faveur de l'interopérabilité des grandes plateformes, afin de fluidifier le passage des utilisateurs de l'une à l'autre ; ceux-ci pourront réellement choisir les plateformes dont les politiques de modération des contenus leur conviennent le mieux. Mes chers collègues, une nouvelle fois, la commission des lois a tenté de tenir une délicate ligne de crête entre, d'une part, la protection des victimes de haine et, d'autre part, la protection de la liberté d'expression telle qu'elle est pratiquée dans notre pays- il ne faut sacrifier ni

par le Gouvernement, après un événement médiatique lié à la campagne électorale parisienne et le vote à l'unanimité d'une proposition de loi visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace. vote éclairent singulièrement les limites du présent texte, sa probable inefficience, mais aussi les limitations qu'il pourrait imposer à la liberté d'expression. Dans l'affaire parisienne que j'ai évoquée, un réseau, prétendument social, a contribué à la propagation massive d'images rendues publiques sur un site internet hébergé par un opérateur étranger. images n'auraient sans doute pas connu pareille notoriété sans l'amplification offerte par ce réseau, qui a joué le rôle de chambre d'écho. Leur diffusion est sévèrement punie par la loi, mais leur signalement par la médiation malfaisante de ce réseau social échappe aux dispositions de la présente proposition de loi. Pourtant, à n'en pas douter, cette plateforme a capté ces pulsions scoptophiles pour son profit, en suscitant la curiosité de ses usagers. Il est regrettable qu'un député ait pu participer à l'animation de cet étalage obscène. En l'occurrence et de manière générale, les plateformes sont les complices intéressés de la propagation de ces contenus illicites, qui constituent la matière de cette économie de l'attention sur laquelle elles ont bâti leur empire monopolistique. Il est donc vain, naïf vain, naïf et risqué de leur confier la régulation des flux qui font leur fortune. Lors du débat sur la proposition de loi visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace, défendue par notre collègue Sophie Primas, à mon interpellation sur la nécessité d'agir sur les causes structurelles de la suprématie néfaste des Gafam, vous m'aviez répondu, monsieur le secrétaire d'État : « Ce qu'il faut, c'est mettre en place une régulation structurante, qui soit intrusive dans le de ces

les effets pernicieux de cette économie de l'attention, mais encore elle conforte le contrôle des Gafam sur internet en leur attribuant des pouvoirs de police, de censure et de régulation dont ils vont certainement se saisir avec beaucoup plus d'efficacité que le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui a pourtant la mission de les surveiller. De façon quasi unanime, juristes et défenseurs de la liberté d'expression et de la neutralité de l'internet vous ont mis en garde contre cette dépossession des pouvoirs régaliens de l'État au profit d'entités supranationales qui contestent ses lois. Pis, en obligeant les plateformes à retirer de façon presque immédiate les contenus susceptibles d'être illicites, le Gouvernement les incite à développer des outils d'analyse des comportements de leurs usagers, afin de les rejeter préventivement, ou à élaborer, en toute opacité, leurs propres critères de censure qu'elles activeront de manière automatique, sans aucune possibilité de recours. Le blocage du site du Syndicat des avocats de France est l'une des dernières manifestations du pouvoir absolu et discrétionnaire accaparé par les plateformes. La prise de contrôle de l'internet et la capacité de celles-ci de maîtriser, par leurs choix, une partie du débat public constituent un véritable danger pour notre démocratie. Le processus électoral en cours aux États-Unis nous en donne malheureusement, de nouveau, des exemples très inquiétants. Selon la presse américaine, 30 000 internautes reçoivent chaque minute une publicité politique du candidat démocrate ancien maire de New York. Comment nous garantir, monsieur le secrétaire d'État, qu'il ne serait pas possible à un candidat de mettre en oeuvre, en France, des pratiques similaires ? Hannah Arendt pensait que l'on pouvait lutter contre les systèmes totalitaires en s'opposant aussi à leurs technologies. Adaptant cet objectif au temps présent, Kate Crawford nous exhorte à défendre des règles éthiques de collecte des données. Je la cite pour conclure : « Nous sommes dans une course à l'extraction de données, et c'est cette culture qu'il faut changer ! ». La parole

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, depuis la première lecture de ce texte, il y a deux mois, la situation a changé. Une commission mixte paritaire a eu lieu, puis une nouvelle lecture à l'Assemblée nationale ; enfin, ont éclaté les affaires Mila et Pavlenski. Je commencerai par la n'ait pas été conclusive, elle a permis de rapprocher les points de vue de l'Assemblée nationale et du Sénat. Dans sa nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a tenu compte de notre contribution sur le renforcement des sanctions financières et sur l'obligation de transparence des vendeurs d'espaces publicitaires et des annonceurs. Elle nous a suivis en plaçant l'observatoire de la haine en ligne sous la tutelle du CSA et en reconnaissant la nécessité de renforcer la prévention en milieu scolaire. Il ne reste qu'une divergence majeure, et, malheureusement, elle porte sur le coeur du texte initial. Le Sénat a supprimé le délit de non-retrait des contenus haineux dans les vingt-quatre heures, qui constitue la mesure phare du texte, celle qu'attendent les victimes des contenus haineux et les associations qui les défendent. J'ai plaidé sans succès, en première lecture, pour que nous conservions cet article. La commission des lois n'étant pas de mon avis, la tâche était surhumaine. Voltaire disait qu'il est dangereux d'avoir raison quand le Gouvernement a tort ; je dis qu'il est délicat d'avoir raison quand la commission a tort Car je crois que la commission a tort. Je ne me fais guère d'illusion sur le succès de ma nouvelle tentative, mais je compte bien défendre ma conviction jusqu'au bout, et c'est là qu'intervient le deuxième changement de situation que j'évoquais pour commencer : les affaires Mila et Pavlenski sont passées par là. Jusqu'alors, nous avions tous entendu parler de la haine sur les réseaux antisociaux et sur la nécessité de la combattre. Mais, pour beaucoup de nos collègues, cette notion restait virtuelle, soit parce qu'ils ne participent pas à ces réseaux, soit parce qu'ils n'ont pas été personnellement victimes des injures, des menaces ou du racisme qui y sont quotidiennement déversés. L'affaire Mila, médiatisée dans tous ses détails et dans toute son horreur, a permis à la France entière de prendre la mesure du fléau

Il est grand temps de réguler les torrents de boue [ ...] La liberté d'expression doit s'arrêter aux frontières de la vie privée que chaque citoyen est en droit d'exiger. » Ces paroles méritent, me

Supprimant cette sanction, le texte du Sénat ne sera qu'une énième version des voeux pieux que sont les lois existantes, avec le même résultat, c'est-à-dire rien ! Le Sénat n'aura pas les mains sales, parce qu'il n'aura pas de mains. Pourquoi le Sénat ne veut-il pas avoir les mains sales ? Parce qu'il craint que ce texte ne porte atteinte à la sacro-sainte liberté d'expression. Si tel était le cas, je serais le premier à m'y opposer ; je vais donc expliquer pourquoi cette crainte relève d'une erreur d'analyse. Il faut d'abord le dire clairement : la haine, les menaces, le racisme, l'injure, le sexisme, l'homophobie ne relèvent pas de la liberté d'expression ; ce sont des délits. On nous explique qu'en donnant aux plateformes la responsabilité de faire cesser ces délits nous privatiserions la censure, nous leur confierions ce qui doit être confié au juge. Comment peut-on soutenir cela, alors que le mécanisme est basé exactement sur le même principe que celui qui s'applique à la presse depuis 1881 ? La loi de 1881 précise que la presse n'a pas le droit de livrer de contenus haineux, de diffamer ou d'injurier. La presse s'y conforme depuis toujours, elle contrôle ses contenus et personne n'a jamais dit qu'on lui confiait le rôle du juge. L'erreur de raisonnement consiste à distinguer les éditeurs, c'est-à-dire la presse, et les hébergeurs, autrement dit les plateformes, alors qu'ils ont un point commun ce sont des diffuseurs. C'est la diffusion qui compte en la matière. De ce point de vue, plateformes et presse ont les mêmes responsabilités. La liberté d'expression, ce n'est pas de diffuser de la haine, de la violence, des appels au meurtre ou au viol, ce n'est pas d'empêcher les autres de s'exprimer par du harcèlement, des attaques massives ou des menaces. En confondant ces délits avec la liberté d'expression, ce ne sont pas les victimes que l'on défend, mais ce sont les agresseurs. Ce texte vise seulement à appliquer les mêmes règles, les règles de 1881, à la presse et à internet. Personne ne peut affirmer qu'en l'adoptant nous allons triompher des « torrents de boue » dont parle Gérard Larcher tant le problème est grave. Mais s'il n'est pas adopté, je suis certain que la partie est perdue d'avance.

Mes convictions n'ont pas évolué sur cette proposition de loi, que nous examinons aujourd'hui à la suite de l'échec de la commission mixte paritaire. Clairement, le Sénat a jugé que les dispositions contenues à l'article 1 présentaient des risques non négligeables et non évalués pour la liberté d'expression. Je le maintiens : ce n'est pas à nos sociétés de s'adapter aux plateformes, mais c'est aux plateformes de respecter nos valeurs les plus fondamentales. Si cet échec est regrettable, il était cependant

et ceux qui en sont victimes. Il serait cependant trop facile et trompeur d'opposer un Sénat conservateur insensible à cette problématique à un gouvernement et à une majorité animés de bons sentiments, et porteurs de solutions innovantes et efficaces. Très c'est pourquoi cet échec était également prévisible -, vous avez privilégié une procédure accélérée qui n'a pas permis de faire converger les approches. Contrairement à ce que suggère l'Assemblée nationale, l'avis du Conseil d'État est loin d'être positif et celui de la Commission européenne est franchement critique. Hier, j'assistais encore à une réunion de travail à l'ambassade du Canada

Je regrette véritablement que, sur un sujet aussi important, nous n'ayons pas pu prendre ensemble un peu de hauteur. Plutôt que de vous lancer dans cette série de propositions de loi tentant de bricoler des solutions, il aurait mieux valu aborder le sujet de manière systémique. Nos amis britanniques, par exemple, ont décidé de traiter la question dans sa globalité, en évitant l'accumulation de textes puzzles. Ils ont ainsi annoncé mercredi dernier le renforcement des pouvoirs de l'autorité régulatrice des télécommunications au Royaume-Uni, (Ofcom), qui rassemble l'équivalent

est d'autant plus regrettable que d'autres pays nous observent et prennent souvent exemple sur notre législation. Il est aussi question de l'impulsion que souhaite donner la France et des réponses qu'elle veut voir apporter sur le plan international à cet enjeu du XXI siècle. Il convient d'évoquer deux autres points, illustrés par l'actualité récente et à venir. Tout d'abord, d'abord, la question des moyens reste entièrement posée. Notez, monsieur le secrétaire d'État, que sur les dispositions de l'article 4, qui élargissent les prérogatives du CSA dans le cadre d'un contrôle systémique, nos positions étaient très proches de celles de l'Assemblée nationale, qui a d'ailleurs conservé les

encore, tout est question de volonté et de moyens. C'est un sujet qui m'est cher puisque dès 2011 je faisais inscrire dans le code de l'éducation la nécessaire sensibilisation aux potentiels d'internet, mais aussi à ses risques d'internet, mais aussi à ses risques et à la nécessité de maîtriser son image. Des exemples récents et malheureux montrent à quel point même des personnes que l'on pourrait croire très bien informées peuvent se laisser piéger ! Nombreuses sont les victimes de l'attrait irrésistible de la communication instantanée, gratuite et virtuelle conçue pour nous faire oublier que le monde numérique est tout aussi sauvage et impitoyable que le monde réel. Dans ce contexte, monsieur le secrétaire d'État, je ne peux une nouvelle fois que vous d'urgence et concrètement la montée en compétence numérique de tous, à commencer par celle des décideurs. J'ai été effrayée d'entendre à la radio le nouveau ministre des solidarités et de la santé, parlant de la capacité de réactivité de la Chine face au coronavirus qui a pris « des mesures de confinement très rapidement », préciser : « Je ne suis pas sûr qu'il serait possible de réaliser ça dans un pays où les réseaux sociaux seraient ouverts » ! Protection de la vie privée, manipulation des données et de l'information, contenus haineux, concurrence déloyale, abus de position dominante : c'est l'écosystème numérique que nous avons laissé béatement se développer qui pose fondamentalement problème, c'est l'hyperpuissance de ces oligopoles aux mains desquels toute notre vie est en passe de se trouver piégée. Excellent ! L'entrepreneur Tariq Krim n'hésite pas à affirmer que « les grandes plateformes sont la de la pensée

permettre de passer à une nouvelle étape de développement basée sur des principes respectueux de nos libertés ? Comme Tariq Krim, je crois au progrès, à un modèle éthique et durable

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de vous présenter des excuses : je supplée aujourd'hui Marie-Pierre de la Gontrie, qui connaît mieux que moi les enjeux de ce texte. Cependant, comme parlementaire attaché au numérique et à la liberté d'expression, j'essaierai de lui faire honneur Depuis la première lecture de ce texte par notre assemblée en décembre dernier, l'actualité est venue nous rappeler très régulièrement combien internet était un formidable outil d'expression et de communication, mais également un espace où se propagent les attaques, la haine, les menaces ou l'incitation à la violence. Le cas de Mila, cette jeune fille de 16 ans attaquée et menacée pour avoir exprimé des opinions sur une religion, qui a fait couler beaucoup d'encre, en est un exemple. Sur un sujet aussi important que la lutte contre les contenus haineux sur internet, nous ne pouvons que regretter l'échec de la commission mixte paritaire et l'absence de consensus. L'objectif qui sous-tend cette proposition de loi est partagé. Nous en convenons tous. Mais les désaccords sur les moyens d'y parvenir ont persisté. Pour sa part, le groupe socialiste et républicain aborde cette seconde lecture comme il l'a toujours fait, avec un esprit de responsabilité. Nous sommes convaincus de la nécessité de faire évoluer l'arsenal législatif pour répondre à la prolifération de la haine sur internet, c'est-à-dire à l'expression et à la diffusion de cette

Oui, nous avons le devoir de sanctionner les auteurs de contenus haineux et de responsabiliser les plateformes. Oui, nous devons trouver les moyens de réagir vite pour contenir la viralité de ces contenus, car il s'agit avant tout de protéger les victimes. la recherche d'une efficacité toute relative dans cette lutte ne saurait en aucun cas justifier de recourir à des moyens potentiellement attentatoires aux libertés publiques. Tel était et demeure encore aujourd'hui notre fil conducteur pour aborder ce débat. Le texte qui nous est soumis n'a cessé d'évoluer depuis sa première version adoptée par l'Assemblée nationale en juillet dernier, preuve s'il en était de l'intérêt du débat parlementaire et de la navette entre les deux chambres. Pour autant, les réserves qu'il suscite sont toujours aussi nombreuses et continuent de nous interpeller. Dans une démarche constructive, nous avons déposé plusieurs amendements qui visent à réaffirmer les principes essentiels pour notre groupe et à améliorer un texte qui reste encore imparfait. Tout d'abord, nous proposons d'exclure explicitement la presse du champ de cette proposition de loi. Les auteurs du texte n'ont pas jugé nécessaire de distinguer les organes de presse parmi les auteurs potentiels de contenus. Nous avions soulevé ce point en première lecture et avions été stupéfaits d'entendre en séance la garde des sceaux affirmer qu'il était difficile d'accorder un traitement spécifique aux entreprises de presse. Or ne pas exclure explicitement la presse du champ d'application de la future loi introduirait un flou dangereux et rendrait de fait possible le retrait en par un opérateur de plateforme, des propos émanant d'un organe de presse. Nous sommes, je le pense, toutes et tous, ici, attachés à la liberté de la presse, essentielle à la démocratie. Il nous semble primordial de le rappeler.

Ce sujet a d'ailleurs constitué le principal point d'achoppement entre les deux chambres. En commission, le Sénat a, de nouveau, fait le choix de rejeter l'instauration de ce délit. Nous regrettons que les propositions que nous avions faites, et qui visaient à dépasser cette problématique, aient été rejetées en première lecture. Nous avons voulu les formuler de nouveau. Il s'agit d'instaurer une obligation de retrait ou de blocage à titre provisoire d'un contenu haineux notifié, sous un délai de vingt-quatre heures, jusqu'à sa validation par le tribunal judiciaire statuant en référé. Cette proposition permettait de concilier l'efficacité de la lutte contre la haine en ligne et le respect du rôle de la justice, à qui il revient de se prononcer et de trancher sur la possibilité de limiter la liberté d'expression. Enfin, d'autres points nous semblent encore nécessiter des améliorations, notamment s'agissant de la supervision opérée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les opérateurs de plateforme en ligne en matière de lutte contre les contenus haineux. Nous souhaitons sur ce sujet faire quelques propositions qui nous semblent importantes pour renforcer l'action du Conseil, notamment en matière de contrôle des algorithmes. Nous y reviendrons au cours de la séance.

force est de le constater, la réalité nous a une nouvelle fois rattrapés lors de l'examen de cette proposition de loi visant à lutter contre la haine en ligne. Encore, la haine frappe en ligne et toujours sous le sceau de l'anonymat. Mais s'il est nécessaire de légiférer sur ce sujet, il faut le faire de manière dépassionnée et en visant un texte ayant le plus d'effectivité possible dès son entrée en vigueur. Il faut aussi prendre son temps, et c'est sans doute ce qui nous a manqué pour parvenir à un texte de compromis avec l'Assemblée nationale.

L'autre point d'achoppement est le fait d'intégrer les moteurs de recherche dans le champ de la proposition de loi. L'Assemblée nationale s'y évertue bien que ceux-ci ne jouent pas un rôle majeur dans la diffusion des propos. Loin de nous rassurer, les apports de nos collègues députés en deuxième lecture ont suscité une certaine incompréhension. L'ajout à l'article 1 d'une disposition visant à créer une obligation de suppression en une heure des contenus à caractère terroriste

laquelle je tiens à saluer une nouvelle fois le travail effectué par le rapporteur, qui a permis le retour à un texte équilibré. Le rétablissement à l'article 1 de l'abrogation de la sanction à l'encontre des hébergeurs ne supprimant pas les contenus haineux s'inscrit dans la droite ligne des propos que nous avons pu tenir. À l'article 2, la proportionnalité des obligations de moyens renforcées mises à la charge des grands opérateurs de plateforme prend en compte les différences entre les opérateurs. En effet, selon leur taille et leurs moyens, ceux-ci ne disposent pas de la même force de frappe pour lutter contre les propos haineux. Il était donc nécessaire de s'adapter, au risque de renforcer les plateformes déjà hégémoniques et de pénaliser les plateformes Je soulignerai enfin les apports de la commission de la culture, notamment à l'article 4, qui permettent de donner davantage de prérogatives au CSA pour établir des recommandations concernant les obligations de moyens et de diligence des opérateurs en ligne. Sont aussi à mettre à son crédit les différentes dispositions visant à lutter contre la viralité et à favoriser l'interopérabilité, enjeux sur lesquels j'avais mis l'accent en première lecture. Tous ces éléments nous permettent d'avoir un texte qui, s'il n'est certes pas parfait, comme je l'ai déjà souligné, nous met en accord avec nos engagements européens. Je regrette d'autant plus nos désaccords avec l'Assemblée nationale que sur bon nombre de sujets nous sommes en phase, notamment sur la régulation des grandes plateformes, sur l'interdiction de la surveillance généralisée ou sur le contrôle des algorithmes. Nous sommes également d'accord sur la nécessaire prévention quant à la haine en ligne. Car trop souvent l'absence de suivi, d'écoute et de sensibilisation conduit au drame chez les publics les plus sensibles- je pense aux enfants. La formation des enseignants et le renforcement des sanctions pour les mineurs étaient donc nécessaires.

ensuite, parce qu'en parallèle la législation bruxelloise évolue, avec l'obligation pour les pays membres de transposer la directive Service des médias audiovisuels (SMA), qui fixe le socle de règles communes pour les plateformes de partage de vidéos, les réseaux sociaux et les plateformes de diffusion en direct.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, internet est un espace de coexistence sociale à nul autre pareil, une sorte de nébuleuse où nos libertés fondamentales se contorsionnent sous l'effet de la viralité, où le laissez-faire algorithmique prospère sur fond de juridique, où la violence sociale opère à visage masqué sous couvert d'anonymat. Ce sont autant d'éléments à la lecture desquels le champ de l'économie numérique met à l'épreuve la boîte à outils du législateur. Le législateur, justement, se doit de rappeler aux espaces en ligne, aussi vertueux soient-ils, que le droit, sur ce terrain-là aussi, a sa place. À plus forte raison encore lorsque les pratiques constatées, ici et là, suscitent l'indignation légitime d'un grand nombre de nos concitoyens. Comme le suggère le titre de cette proposition de loi, internet n'a pas fait, hélas !, rempart aux atteintes à la dignité de la personne humaine. Pis encore, il a eu pour effet d'en exacerber les traits les plus révoltants.

car aujourd'hui le législateur répond. Je commencerai par citer les éléments qui nous rassemblent. D'abord, une logique de responsabilisation des opérateurs de plateforme en ligne par un dispositif de régulation administrative, assurée par le CSA, permettra à ces acteurs de déployer tous les moyens nécessaires aux fins de lutter contre la haine sur internet, en se conformant à leurs obligations de moyens, de coopération et de transparence dans la modération de leurs contenus. Ensuite, face à des facilités de sur-censure, il a été utilement reconnu au CSA la faculté de sanctionner sur internet des comportements de retrait excessif. A également été renforcée la lutte contre les sites miroirs, redoutable fléau dans la lutte contre les contenus haineux. Quant aux auteurs de ces contenus, ils seront dorénavant mieux poursuivis, grâce à un parquet numérique spécialisé, qui pourra être saisi au moyen du système de plainte en ligne institué dans le cadre de la loi de programmation et de réforme pour la justice. Malgré ces avancées importantes auxquelles ont contribué nos deux assemblées, des points de divergence demeurent. La commission mixte paritaire a ainsi entériné deux désaccords de fond, qui persistent après l'examen du texte en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale et en commission des lois au Sénat. Le premier concerne le délai couperet de Le Sénat l'a retiré du texte au motif d'une crainte de censure, de « surblocage » et de contournement de l'autorité judiciaire. Mais le délit autonome de refus de retrait avait, bien au contraire, pour objet de redonner toute sa place à l'autorité judiciaire, seule compétente pour apprécier les limites susceptibles d'être portées à la liberté d'expression. Ce délit de non-retrait en vingt-quatre heures offrait, par ailleurs, une portée effective aux dispositions actuelles de la directive e-commerce et de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Son objet était non pas de contrevenir à la liberté d'expression, mais bien au contraire de lutter efficacement sur internet contre ce qui dans le domaine public, au quotidien, n'est ni permis ni toléré. C'est pourquoi mon groupe y était et y demeure favorable. Autre pierre d'achoppement importante, la délimitation du champ des opérateurs visés par ce dispositif législatif. Le Sénat a décidé d'exclure les moteurs de recherche, tout en permettant au CSA d'attraire dans le champ de sa régulation les sites internet qui acquièrent en France un rôle significatif, dans un « en même temps » d'une cohérence discutable. D'autant que ces moteurs de recherche avaient été intégrés au champ d'application de l'article 1 sur préconisation du Conseil d'État, afin non seulement de tenir compte de leur rôle décisif dans l'exposition des contenus publics en ligne, mais aussi de ne pas contrevenir aux principes d'égalité et de non-discrimination. Enfin, outre ces mesures phares, comment ne pas regretter que notre dispositif de transparence des régies publicitaires ait vu son contenu assoupli et sa portée effective réduite à l'Assemblée nationale ? Fort heureusement, l'opportunité de ce mécanisme de démonétisation des plateformes propagatrices de contenus haineux n'est pas, déjà, de l'histoire ancienne. Le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique nous permettra d'en débattre de nouveau. pour toutes ces raisons, et en l'état du texte, le groupe La République En Marche s'abstiendra, tout en espérant que le, projet européen sur la régulation des contenus en ligne destiné à adapter la directive e-commerce aux enjeux présents, permettra de conforter juridiquement nos travaux.

exposé comment ce risque de sur-censure était accentué par le fait que la plupart des plateformes et des opérateurs étaient étrangers-

Or je découvre qu'une parlementaire qui est en pointe en matière de lutte contre les contenus haineux, et donc racistes, estime que tel n'est pas cas ! Mes chers collègues, je vous avais fait part de mes craintes de voir la censure confiée à des pays étrangers qui n'ont pas la même sensibilité que nous sur ce sujet.

mais pour essayer d'apporter des solutions sérieuses, efficaces, respectueuses de la Constitution et conformes à nos engagements européens, à des problèmes réels bien observés et sérieusement analysés. C'est pourquoi nous avons certainement un temps de retard sur les nouvelles générations politiques, qui semblent avoir fait de la communication l'alpha et l'oméga de l'action publique. Chacun d'entre nous, monsieur le secrétaire d'État chargé du numérique, a jugé à sa juste valeur votre propos introductif. Nous avons mesuré son élégance, apprécié son esprit de nuance, constaté le sens de la mesure qui l'a inspiré. Nous avons également relevé votre très grand souci d'objectivité et le respect que vous avez exprimé pour le travail de notre assemblée. Mais je veux vous dire que nous ne pouvons pas faire de bonnes lois avec des voeux pieux et des formules juridiques approximatives, qui n'ont aucune chance de modifier en quoi que ce soit les pratiques. Vous avez cru judicieux de citer l'affaire Griveaux. Ce n'est pas nous qui en parlons, car c'est hors de propos

Cela n'a rien à voir avec le traitement de la haine sur internet ! Le président du Sénat a heureusement réagi, au nom de notre assemblée, en disant qu'il fallait réguler les « torrents de boue » qui se déversent sur internet. Il serait peut-être temps, en effet, que le Gouvernement s'en occupe réellement ! J'ajoute que s'il y a une leçon à tirer de cet épisode tout à fait regrettable, c'est bien qu'il ne faut pas attendre les droits d'une personne sont lésés au degré où elles l'ont été dans cette affaire. Car il n'a fallu que quelques heures à plus de 4 millions d'abonnés aux réseaux sociaux pour visionner

les plateformes à prendre des précautions en censurant des expressions qui s'avéreraient finalement ne pas avoir de contenu ne pas avoir de contenu réellement haineux. Voilà la raison fondamentale pour laquelle vous vous êtes orienté, faisant suite, il est vrai, à la proposition de loi déposée par une parlementaire de votre majorité, vers une fausse solution, une fausse sécurité

que je constate la persévérance dans l'erreur de ce gouvernement, alors que le Sénat ne demandait pas mieux que de l'aider à mettre en place un dispositif constitutionnel, conforme au droit européen et efficace

étendu aux publications audiovisuelles et en ligne. Une véritable ambiguïté subsiste sur le champ d'application du texte dont nous débattons, et nous préférons qu'elle soit expressément levée. Il serait Il serait invraisemblable que la responsabilité juridique des éditeurs de presse, voire des journalistes, puisse éventuellement être retenue sur la base des dispositions applicables aux opérateurs de plateformes, et qu'ils soient tenus à de nouvelles obligations et passibles de nouveaux types de sanctions. Je rappelle que la responsabilité juridique des éditeurs de presse quant aux contenus qu'ils publient est déjà engagée par la loi du 29 juillet 1881, dans ses articles 23, 24 et 24 , qui soumet à sanction les cas de publication de propos injurieux,

les éditeurs de presse en ligne sont déjà responsables de la modération des commentaires en ligne. Les lois restreignant actuellement la liberté d'expression et celle de la presse- liberté pourtant érigée en principe à valeur constitutionnelle -sont dans l'air du temps. Nous avons déjà alerté il y a un an, lors des débats préalables à son adoption, sur les dommages collatéraux pour la presse que pourrait contenir la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information. Les conditions d'exercice de la presse sont de plus en plus précaires et difficiles, tant financièrement parlant qu'en termes de conditions de travail, ou encore sur le plan déontologique. La période est à la censure accrue, qui menace d'induire une autocensure. N'aggravons ni les conditions d'exercice des journalistes ni celles des éditeurs de presse. La liberté d'expression et celle de la presse constituent l'un des principaux fondements de la démocratie. je vous demande de bien vouloir adopter notre amendement, qui garantira à la presse de continuer d'informer dans un régime de responsabilité respectueux de la liberté.

L'amendement présenté par M. Durain a pour objet d'exclure la presse du champ d'application de la présente proposition de loi. Je le redis, nous avions évoqué ce sujet en première lecture, et nous nous souvenons tous que la réponse de la garde des sceaux nous avait plongés dans une certaine perplexité, pour dire le moins. Il s'agit manifestement, et c'est ainsi que je l'entends, monsieur Durain, d'un amendement d'appel, qui devrait cette fois-ci, puisque la garde des sceaux n'est pas là- fort heureusement ! -, donner au Gouvernement l'occasion de corriger le tir et de rassurer les éditeurs de presse en ligne. Pour ma part, j'avais donné une explication qui avait satisfait tout le monde jusqu'à ce que la garde des sceaux prenne la parole Sur le fond, et je reprends mon rôle de rapporteur, la réponse n'a toujours pas changé : cet amendement n'est, à mon sens, pas réellement utile et pas opérant juridiquement. Je vais m'en expliquer, peut-être pour la dernière fois, en tout cas je l'espère. D'abord, n'oublions pas que le régime de responsabilité des éditeurs n'est absolument pas modifié par la présente proposition de loi. effet, ce texte ne concernera que les hébergeurs, et uniquement les plus grands d'entre eux, ceux qui dépassent un seuil de connexion. Les contenus publiés en ligne par les entreprises de presse qui ont juridiquement le statut d'éditeur n'étant pas visés pas visés par ce texte, leur exclusion me semble donc inutile. Du reste, la rédaction de cet amendement ne me paraît pas opérante juridiquement, pour deux raisons. La LCEN recourt non pas à la notion de presse à proprement parler, mais aux termes plus précis d'éditeur et d'hébergeur, définis par la loi et, surtout, par la jurisprudence. L'exclusion générale à instaurer le présent amendement se fonde sur la finalité économique de l'activité poursuivie- la presse -et non sur la nature technique de la prestation- hébergeur, éditeur. Cette disposition poserait probablement des problèmes d'égalité devant la loi. il peut arriver que des entreprises de presse soient aussi responsables, comme hébergeurs, d'une partie accessoire de leur activité, si elles ont des forums de lecteurs ou ouvrent des zones de commentaires en ligne. On ne peut donc pas les exclure de façon aussi générale de l'application de la loi. Dans ces conditions, monsieur Durain, je vous demande

le 15 janvier dernier, lors de ses voeux à la presse, M. le Président de la République indiquait que, « en France, la liberté de blasphème est protégée. » Il ajoutait : « nous ne nous lasserons jamais de défendre la liberté d'expression, dans toute sa plénitude.

... Surtout, le parquet de Vienne décida d'ouvrir deux enquêtes : l'une sur les menaces de mort à l'égard de Mila et l'autre pour déterminer si les propos de l'adolescente relevaient éventuellement de la provocation à la haine raciale alors même, je le rappelle, qu'aucune plainte n'avait été déposée.

Encore une fois, les propos de Mila n'étaient pas contraires à la loi ; en revanche, votre faux parallélisme- le déclenchement d'une action publique à l'égard des deux protagonistes -affaiblit, me semble-t-il, vos propos et votre volonté affirmée de réguler la haine. Tout cela est profondément regrettable.

de la création du délit de non-retrait, en vingt-quatre heures, des contenus haineux notifiés aux grandes plateformes, figurant à l'article 1. À ce stade du débat, la majorité gouvernementale comme la majorité sénatoriale maintiennent la position qu'elles ont adoptée en première lecture, situation qui a conduit à l'échec de la commission mixte paritaire réunie le mercredi 8 janvier dernier. Nous partageons les observations du rapporteur de la commission des lois à l'égard du dispositif adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, lequel risque d'entraîner, par précaution, des sur-retraits de propos licites, mais polémiques. En effet, si un doute subsiste sur la nature du contenu, les opérateurs préféreront le retirer plutôt que de risquer le paiement automatique d'une amende. Pareil dispositif reviendrait à conférer à des entreprises dominantes dans ce secteur une responsabilité exorbitante, s'apparentant à une compétence régalienne, aux dépens de la liberté d'expression. En supprimant de nouveau les mesures contraignantes adoptées par les députés pour les remplacer par de simples obligations de moyens, notre commission des lois parie sur le seul volontarisme des opérateurs à fort trafic, dont on sait que les principales préoccupations reposent avant tout sur des considérations économiques liées à la marchandisation croissante d'internet. Compter sur l'action spontanée d'acteurs dominants dans les services de communication au public en ligne sous le contrôle incitatif du régulateur sera insuffisant pour favoriser l'évolution du droit en vigueur, unanimement considéré comme inadapté. Nous ne pouvons nous résoudre à l'inaction. Pour sortir de cette impasse, nous devons apporter les garanties qui permettraient de satisfaire l'ensemble des acteurs de la société civile et de l'économie du numérique, en réservant à l'autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles et de la liberté d'expression, la place qui lui revient dans le dispositif de contrôle. C'est pourquoi nous proposons que le retrait des contenus haineux notifiés soit provisoire, dans l'attente d'une validation par le juge des référés, seul à même d'assurer l'analyse du contexte du retrait dans un délai raisonnable, pour éviter tout risque de sur-censure. En outre, afin de profiter des apports de la navette entre les deux chambres, nous envisageons de reprendre plusieurs mesures qui nous semblent pertinentes : d'abord, nous pensons qu'il convient de maintenir l'intégration des moteurs de recherche dans le champ d'application du dispositif, en raison de la capacité de ces derniers à accentuer la viralité des contenus haineux sur internet ; ensuite, la suppression de la peine de prison au profit du seul prononcé d'une amende est une solution raisonnable, à conserver dans le dispositif ; enfin, les précisions apportées au caractère intentionnel du délit seront utiles pour responsabiliser davantage les grands opérateurs.

raisons essentielles. D'abord, la saisine du juge des référés serait, d'après le mécanisme que vous proposez, systématique il faudrait le saisir après chaque retrait de contenu, même lorsque l'auteur de ce contenu litigieux ne le conteste pas et même dans les cas d'évidence. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les ordres de grandeur ; pour YouTube, on parle de millions de retraits chaque mois.

le référé obligatoire relèverait uniquement de l'initiative des seuls intermédiaires techniques. La procédure que vous envisagez ne précise pas la place, dans cette instance, de l'auteur du contenu ni de l'auteur de la notification, qui ont, pourtant, les meilleurs arguments à faire valoir devant un juge. Je ne peux pas plus vous suivre à propos de l'inclusion des moteurs de recherche dans le champ du délit, disposition que vous rétablissez tout en omettant, d'ailleurs, de prévoir un référé dans ce cas. Le Sénat les avait exclus, jugeant leur rôle bien moins déterminant que celui des réseaux sociaux dans la propagation de la haine. Surtout, les caractéristiques techniques des moteurs de recherche rendent quasiment impossible de désindexer un seul propos haineux précis- un commentaire ou une image -sur la page d'un média, d'un forum ou d'un site de débat participatif, sans rendre inaccessible ou invisible tout le reste, donc tous les autres contenus, pourtant licites. outre, vous supprimez diverses améliorations de la LCEN, pourtant adoptées par le Sénat- message de substitution, durée de conservation des contenus illicites -, qui nous semblaient au contraire très utiles.

une modalité d'information des auteurs dont les contenus ont été retirés et un rappel des modalités d'appel auxquelles ils ont accès. Nous avons donc atteint là un bon équilibre

Maryvonne Blondin. L'article 1 B ouvre aux associations de protection de l'enfance la possibilité de notifier un contenu haineux dont elles sont saisies par un mineur. Dans ce cadre, l'Assemblée nationale a rendu systématique l'information des représentants légaux dudit mineur. Ce choix témoigne d'une méconnaissance de la réalité du terrain et d'un manque de pragmatisme. la plupart du temps, les mineurs victimes de propos haineux sur les réseaux sociaux ne souhaitent pas que leurs représentants légaux soient informés quand il s'agit de certains aspects de la vie touchant à leur intimité, en particulier dans un contexte de violence. Tout l'intérêt de l'article 1 B repose sur l'intervention d'un tiers de confiance, que constitue une association de protection de l'enfance, afin de favoriser les notifications et d'éviter que les mineurs ne renoncent à signaler tout type de contenu haineux, de peur que cette information ne soit communiquée systématiquement à leurs parents. Loin de nous l'idée de déresponsabiliser les parents, mais nous pensons qu'il faut privilégier l'intérêt de l'enfant, en laissant aux structures associatives, reconnues d'utilité publique, le soin de vérifier les faits, de bien en assurer la qualification et de procéder au signalement des contenus haineux. Elles savent faire ; en effet, fortes de leur expérience en la matière, elles sont reconnues tiers de confiance et ont élaboré, avec les plateformes, des procédures prioritaires, qui assurent une réaction rapide et efficace. Il leur reviendra ensuite de poursuivre l'accompagnement du mineur, en favorisant, autant que possible, l'échange avec les parents ou avec un adulte de confiance.

L'amendement n° 4, que vous venez de défendre au nom du groupe socialiste et républicain, madame Blondin, vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture. Il prévoit une exception à l'information, normalement systématique, des représentants légaux du mineur. Serait ainsi réservé le cas où cela est contraire à l'intérêt de l'enfant. L'information des représentants légaux du mineur ayant saisi l'association est un sujet délicat. Elle doit évidemment être la norme, mais, lors de leurs auditions, les associations de protection de l'enfance sur internet se sont inquiétées de l'absence d'exception à cette information systématique. En effet, les contenus litigieux qui leur sont signalés pour en obtenir le retrait font parfois référence à la vie affective et aux pratiques ou à l'orientation sexuelle, vraie ou supposée, des victimes mineures, qui ne souhaitent pas les voir dévoilées à leurs proches ou, en tout cas, L'absence d'exception à l'obligation d'information systématique des représentants légaux risquait donc de décourager lesdits mineurs de recourir à ces associations pour leur venir en aide. Les députés ont supprimé toute exception et ont rétabli en nouvelle lecture le caractère systématique de l'information des représentants légaux des mineurs. Ils ont précisé que cette information se fait « selon des modalités adaptées à l'intérêt supérieur de l'enfant ». Tout le problème qui se pose aujourd'hui est donc de savoir si cette phrase doit être interprétée comme permettant bien aux associations de différer l'information aussi longtemps que l'intérêt supérieur de l'enfant l'exigera. Par conséquent, je sollicite l'avis du Gouvernement. À défaut d'obtenir des assurances suffisantes sur cette interprétation, je proposerai d'adopter cet amendement et de revenir à la version du Sénat.

On ne peut laisser à l'enfant fragilisé par les propos haineux qu'il a lus la charge de décider de l'information de ses parents. Son réflexe peut être de ne pas les inquiéter ou de ne pas susciter de réaction de leur part, alors que, en réalité, la réaction et l'action des représentants légaux sont nécessaires. Cela ne peut pas non plus relever de l'association, qui ne connaît pas les détails de la dynamique familiale du mineur. Les parents ne peuvent exercer leur mission de protection de leur enfant que s'ils sont pleinement informés de ses agissements. Il faut noter que la proposition de loi a déjà été aménagée pour prévoir que cette information soit faite selon des modalités adaptées à l'intérêt supérieur de l'enfant ». J'ajoute que le droit commun de la protection de l'enfance répond déjà parfaitement à la nécessité de ne pas prévenir les parents

Ainsi, dans l'hypothèse où les parents seraient eux-mêmes identifiés comme une source de danger, l'association peut alors transmettre une information préoccupante ou effectuer un signalement sans information des parents si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. L'objectif de la proposition de loi ne justifie donc pas de remettre en cause l'équilibre délicat, mais satisfaisant, entre la protection des intérêts de l'enfant et la responsabilisation de ses parents qui est préservé dans la rédaction actuelle du texte. Dans ces conditions, j'invite ses auteurs à retirer l'amendement, faute de quoi nous y serons défavorables.

contre la spoliation de leur caisse de retraite voulue par votre gouvernement, dans le cadre du projet de loi portant réforme des retraites, le Syndicat des avocats de France, qui relayait leur lutte, a vu son site Twitter suspendu pendant une journée

De quel droit le compte du Syndicat des avocats de France a-t-il été suspendu ? C'est un acte grave : nous demandons des explications à TwitterFrance ! Il est grand temps de contrôler les plateformes et leurs règles

vise, comme en première lecture, à réintroduire le juge dans le processus de retrait du contenu haineux. En l'espèce, en cas de contre-notification par l'auteur de contenus litigieux retirés, la plateforme devrait obligatoirement les rétablir, à charge pour le notifiant de saisir le juge des référés. Cher collègue, même si je partage l'esprit de cet amendement, je ne peux

Je décèle, en outre, deux problèmes juridiques dans la procédure que vous proposez. Premièrement, concernant l'intérêt pour agir du requérant, une notification de contenu haineux illicite à un hébergeur peut émaner de toute personne sans qu'elle ait à justifier qu'elle est personnellement lésée par ledit contenu.

Je peux le regretter politiquement- d'ailleurs, le Gouvernement, qui a été accusé, n'y est pour rien -, mais je ne peux pas non plus totalement reprocher à Twitter de prôner une utilisation raisonnée et raisonnable. Or nous connaissons tous le problème que pose le. S'agissant de votre amendement, je reprends à mon compte les arguments de M.

probablement inconstitutionnelle. En effet, il est un peu compliqué, dans un espace privé, d'obliger à remettre en ligne des contenus spécifiquement mentionnés comme illégaux dans les conditions générales d'utilisation. On peut le regretter. C'est un problème dont nous avons déjà discuté. Néanmoins, jusqu'à preuve du contraire, Twitter constitue un espace privé, où certaines règles s'appliquent pour éviter des dérives, mais dont les conditions générales d'utilisation s'appliquent également. À cet égard, les retraits de contenus que nous pouvons tous ici considérer comme abusifs- on peut évidemment penser à l'exemple traditionnel de -n'ont rien à voir avec la loi : ils sont liés aux conditions générales d'utilisation de Twitter.

Nous n'en savons rien, parce qu'elle apprécie seule le niveau de ce seuil. Je sais que, pour certaines campagnes publicitaires, la société Twitter a refusé de diffuser des informations gouvernementales, pour les mêmes raisons. Je souscris tout à fait à votre argumentation : Twitter est une société privée, qui agit selon des règles de droit privé, en fonction de ses conditions générales d'utilisation. Le problème essentiel, dont nous ne parvenons pas à débattre avec vous, est que cette société est dans une situation monopolistique sur

Mme Victoire Jasmin. L'objet de cet amendement est de donner au régulateur le soin d'organiser les outils de coopération et de partage d'informations opérateurs pour mieux lutter contre les contenus haineux sur internet. Pour rappel, en première lecture, le Sénat avait prévu que les outils de coopération et le partage d'informations mis en place par les plateformes à la demande du CSA le soient dans un format ouvert et conforme à ses recommandations. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a souhaité ne plus mentionner la nécessité que ces outils soient conformes aux recommandations du CSA, au motif qu'une telle mention serait contradictoire avec le caractère purement incitatif de la mission dévolue au CSA dans ce domaine. Cette modification est regrettable,

à l'article 4, les missions confiées au CSA, afin d'encourager le partage d'informations entre opérateurs pour lutter contre la dissémination de contenus haineux illicites. L'amendement n° 5 rectifié, que vous venez de défendre,

reprendre ! J'ai peur de devoir poursuivre dans cette direction malheureuse, car il nous semble qu'imposer que les outils de coopération et de partage d'informations entre opérateurs soient conformes aux recommandations du CSA est contradictoire avec le caractère purement incitatif de la mission dévolue au CSA dans ce domaine. Il ne nous semble pas souhaitable d'aller au-delà de ce caractère incitatif s'agissant des contenus concernés par cet article.

du secret des affaires. En revanche, la capacité du CSA à obtenir des informations pertinentes des opérateurs concernés par le dispositif de lutte contre les contenus haineux sur internet conditionne l'exercice même de sa mission et, par conséquent, son utilité. utilité. Loin d'être une précision superfétatoire, il nous paraît indispensable que la loi attribue au CSA des prérogatives adaptées

de la publicité susceptible d'y être diffusée. Il prévoyait que les annonceurs devaient publier en ligne et tenir à jour, au moins mensuellement, les informations relatives aux emplacements de diffusion de leurs annonces, communiquées par les vendeurs d'espaces publicitaires.

que les sites faisant l'objet d'une décision de blocage judiciaire ou administratif. La transparence des dépenses publicitaires ne serait donc plus générale, contrairement à l'objectif de responsabilisation du secteur publicitaire, des annonceurs ou des intermédiaires du web. On peut entendre les inquiétudes des annonceurs et prendre en compte la complexité de la chaîne des acteurs de la diffusion publicitaire comme on a entendu les inquiétudes exprimées par les grandes plateformes. Toutefois, il importe d'insister sur la nécessité de lutter contre la publicité sur des sites diffusant des

Dans le dernier état de sa rédaction, la transparence des dépenses publicitaires ne serait plus générale, mais concernerait uniquement les sites faisant l'objet d'une décision de blocage judiciaire ou administrative. Les acteurs de la publicité en ligne seraient destinataires des listes de sites faisant l'objet d'une demande de blocage et devraient alors rendre publique, au moins une fois par an, sur leur site internet, l'existence de ces relations et en faire mention dans leur rapport annuel. Les auteurs de cet amendement souhaitent aller encore plus loin en généralisant cette transparence à tous les acteurs de la publicité en ligne. La commission vous propose d'en rester

laquelle ne doit pas être confondue avec la liberté de déverser des torrents de boue délictueux. Je n'y reviens donc pas. Je voudrais seulement répondre à deux ou trois arguments que j'ai entendus au cours du débat, à commencer par l'argument d'autorité, utilisé depuis longtemps, selon lequel la version initiale du texte serait inconstitutionnelle et inconventionnelle. Le Conseil d'État, que l'on sollicite un peu trop, souligne pourtant que ce délit « ne viendrait que donner une portée effective aux dispositions actuelles de la directive e-commerce » et de la loi pour la confiance dans l'économie numérique et « ne soulèverait pas de difficulté au regard du droit constitutionnel et des obligations conventionnelles de la France ». Il faut tout de même le dire à un moment ou à un autre. De la même façon, en ce qui concerne la non-conformité au droit européen, je rappelle que la loi allemande, qui prévoit le même délit et va beaucoup plus loin que la loi française, a fait l'objet des mêmes critiques, mais n'a subi aucune censure de la part des instances européennes.

dealers. Tout l'écosystème est concerné. Je voudrais terminer sur une réflexion qui pourrait nous rassembler tous. J'entends les critiques expliquant que l'efficacité du texte initial est sujette à caution- l'avenir nous le dira. De la même façon, je reste convaincu que le texte du Sénat ne sera pas opérant. Nous pouvons toutefois nous accorder sur la certitude que le combat contre la dégradation de plus en plus inquiétante de ce magnifique outil que pourrait être internet sera long, difficile et incertain. Il nécessitera beaucoup d'autres propositions et beaucoup d'autres séances comme celle-ci. Arriverons-nous un jour à faire cesser les deux menaces fondamentales auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui : la diffusion généralisée de la haine et la déstabilisation inquiétante de notre démocratie ? La réponse précise, nette et définitive à cette question est : « Dieu seul le sait », mais cela ne doit pas nous empêcher de tenter ensemble de progresser.

de loi, conforme à ses exigences en matière de respect des libertés publiques. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions des commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 et du projet de loi modifiant la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution et prorogeant le mandat des membres de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le 4 février dernier, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur les projets de loi relatifs à l'application de l'article 13 de la Constitution. L'examen de ces deux textes s'est toutefois avéré plus compliqué que prévu. Initialement, le Gouvernement les présentait comme un travail d'actualisation, voire de coordination, concernant la liste des nominations soumises à l'avis préalable des commissions parlementaires. Il fallait, par exemple,

Sur le plan technique, ce travail de coordination n'était d'ailleurs pas abouti et nous avons dû ajouter des dispositions concernant Bpifrance et l'Autorité Rapidement, nous avons constaté que ces deux textes soulevaient un problème de méthode : nous sommes en effet invités à tirer les conséquences de trois ordonnances qui n'ont pas encore été ratifiées. Je pense notamment à l'ordonnance du 3 juin 2019, qui réorganise de fond en comble la SNCF : plus de huit mois plus tard et malgré nos nombreuses relances, le Gouvernement ne nous a communiqué aucun calendrier de ratification. De même pour l'ordonnance du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, dont chacun connaît les enjeux financiers telle situation me paraît profondément regrettable pour le Parlement et contraire à l'esprit de l'article 38 de la Constitution, qui prévoit la ratification expresse des ordonnances. les projets de loi adoptés en conseil des ministres auraient conduit à un recul, même léger, du contrôle parlementaire sur les nominations aux emplois publics, ce que le Sénat n'a pas pu accepter. Tout au long des débats, nous avons rappelé notre attachement à la procédure prévue par l'article 13 de la Constitution. Créée par la révision constitutionnelle de 2008, elle permet au Parlement de « bloquer » une nomination du Président de la République lorsque l'addition des votes négatifs dans les commissions compétentes représente, au total, au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés. C'est ce que nous appelons les « trois cinquièmes négatifs La procédure de l'article 13 de la Constitution permet ainsi d'écarter des candidatures de complaisance et de renforcer la transparence des nominations, notamment grâce à l'audition des candidats pressentis. Elle mériterait toutefois d'être renforcée, par exemple en modifiant les règles de majorité. Je rappelle que, depuis 2008, le Parlement n'a jamais mis en oeuvre son pouvoir de veto sur les nominations du Président de la République. Il a failli le faire en décembre 2019 pour le directeur général de l'Office national des forêts (ONF), à une voix près. Dès la première lecture, nous avons proposé d'utiliser ce vecteur législatif pour étendre le périmètre des nominations soumises à l'avis préalable du Parlement. Le Gouvernement s'est longtemps opposé à cette volonté de conforter le contrôle parlementaire, ce que nous regrettons. Il n'a toutefois pas été suivi par la commission mixte paritaire, qui a conservé une grande partie des apports du Sénat. Je souhaite d'ailleurs remercier le rapporteur de l'Assemblée nationale, Christophe Euzet, pour son écoute et sa recherche d'un consensus entre les deux chambres. le Parlement sera désormais consulté sur la nomination du président de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Il s'agit d'une revendication ancienne du Sénat, longtemps défendue par notre ancien collègue Jacques Mézard.

Fidèles au rapport rédigé en 2014 par Jean-Jacques Hyest et Corinne Bouchoux, nous pensons au contraire que la CADA joue un rôle fondamental pour garantir les droits des citoyens, alors que la demande d'accès aux documents administratifs n'a jamais été aussi forte. Le Conseil constitutionnel l'a d'ailleurs reconnu dans sa décision du 23 octobre 2014 sur l'accès aux documents administratifs en Polynésie française. Je regrette également que le Gouvernement soit resté muet sur les difficultés rencontrées par cette autorité administrative indépendante. Je rappelle que le « stock » d'affaires de la CADA dépasse aujourd'hui les 1 800 dossiers. Son délai moyen de traitement dépasse les quatre mois, alors que la loi prévoit un délai théorique d'un mois. Une fois sa décision rendue, les citoyens doivent encore attendre deux mois pour obtenir une réponse de l'administration et, le cas échéant, pour se porter devant le tribunal administratif. C'est un vrai labyrinthe, qui fragilise, au bout du compte, le droit d'accès aux documents administratifs. l'initiative de notre collègue Jean-Yves Leconte, le Parlement sera également consulté sur la nomination du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Loin d'assurer une simple mission consultative, l'OFII joue un rôle croissant dans l'accueil des demandeurs d'asile et l'intégration des immigrés en situation irrégulière. Nous nous prononçons déjà sur la nomination du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Il nous semblait donc logique d'y ajouter l'OFII. La commission mixte paritaire a également préservé les apports de l'Assemblée nationale, en ajoutant à la liste des emplois concernés par l'article 13 de la Constitution, d'une part, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et, d'autre part, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Ces deux ajouts me semblent particulièrement judicieux au regard de l'importance de ces deux agences dans la vie économique et sociale de la Nation. Le code de la santé publique prévoyait déjà l'audition de ces dirigeants devant le Parlement. Nous sommes toutefois allés plus loin en prévoyant une capacité de veto en amont de leur nomination. Ce contrôle relèvera de la commission des affaires sociales de chaque assemblée. Au total, 55 emplois publics seraient soumis au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution, soit un de plus qu'aujourd'hui. La privatisation d'Aéroports de Paris pourrait nécessiter de nouveaux ajustements, mais nous n'en sommes pas encore là. Nous n'avions qu'une divergence avec l'Assemblée nationale, concernant la SNCF. Sur l'initiative de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et de son rapporteur pour avis, Didier salue la qualité du travail, le Sénat souhaitait conserver un « droit de regard » sur SNCF Réseau. Il s'agissait ni plus ni moins de maintenir le droit en vigueur, le Parlement étant consulté sur cette nomination depuis 2010. Après avoir auditionné l'Autorité de régulation des transports, nous pensons que SNCF Réseau doit bénéficier de garanties suffisantes d'indépendance, sans remettre en cause la nouvelle architecture du groupe public. En l'état du droit, le compte ne semble pas y être Dans les faits, SNCF Réseau répartira les heures de passage sur les 30 000 kilomètres de voies ferrées entre les sociétés de transport, dont SNCF Voyageurs. Chacun comprend ainsi le caractère sensible de ce dossier. L'Assemblée nationale n'a pas partagé notre point de vue, insistant sur l'« unité managériale » de la SNCF, ce que nous regrettons. Ce débat pourra toutefois se prolonger au moment de la ratification de l'ordonnance du 3 juin 2019 réorganisant la SNCF. À titre subsidiaire, le projet de loi ordinaire vise à proroger le mandat du président de la

au droit commun des autorités administratives indépendantes, doit rester exceptionnelle. Le Sénat sera attentif à sa mise en oeuvre, notamment lors de l'examen du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique. Au bénéfice de ces observations, la commission des lois vous invite, mes chers collègues, à adopter le projet de loi organique et le projet de loi dans leur version issue des travaux de la commission mixte paritaire. Ces textes préservent les principaux apports du Sénat et, donc, le contrôle

et à la prorogation du mandat des membres de la Hadopi, après l'adoption des conclusions de la commission mixte paritaire par l'Assemblée nationale le 11 février dernier. Je suis heureux de constater que les députés et les sénateurs ont réussi à s'accorder sur un texte, qui, je le crois, est de nature à satisfaire toutes les travées. Comme je l'avais exprimé devant vous au mois de décembre dernier, avec ces deux textes, l'intention du Gouvernement est double. Concernant l'article 13 de la Constitution, il s'agit de tirer les conséquences des récentes réformes menées par le Gouvernement- je pense notamment au « paquet ferroviaire » et à la loi Pacte -pour permettre au Parlement d'exercer pleinement son rôle. Concernant la prorogation du mandat des membres de la Hadopi, il s'agit d'éviter d'avoir à nommer de nouveaux membres pour une très courte période et de permettre à l'autorité de continuer à fonctionner convenablement. Lors des premières lectures, le texte a été enrichi par le Sénat et l'Assemblée nationale. Vous êtes parvenus à un accord lors de la commission mixte paritaire, ce dont le Gouvernement se félicite. Je souhaite revenir ici sur deux points qui ont suscité des débats lors des discussions. Le Gouvernement a eu l'occasion, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, d'exprimer ses réserves sur l'ajout du président de la CADA à la liste des emplois concernés par l'alinéa 5 de l'article 13 de la Constitution, les missions de cette commission ne relevant pas du champ d'application de cet article. Sénateurs et députés sont tombés d'accord pour que cette disposition soit maintenue dans le texte final, et nous en prenons donc acte. S'agissant des dispositions relatives à la SNCF, les modifications apportées par votre assemblée n'étaient pas conformes au droit commun des sociétés à participation publique et, tout en comprenant votre souhait d'assurer l'indépendance de SNCF Réseau, par ailleurs garantie par l'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports sur la nomination du directeur général de cette filiale, le Gouvernement ne pouvait pas soutenir la proposition sénatoriale. L'Assemblée nationale est revenue au texte initial du Gouvernement. Nous sommes donc heureux que la commission mixte paritaire ait maintenu les dispositions telles que le Gouvernement les avait proposées en première intention. a également validé les ajouts de l'OFII, de l'ANSM et de l'Anses, issus d'amendements des députés et des sénateurs de différentes sensibilités politiques, à la liste prévue par l'article 13 de la Constitution. Nous avons entendu les remarques exprimées au Sénat et à l'Assemblée nationale concernant les dispositions relatives à la Hadopi. Je tiens à le répéter ici, avec cette mesure, il ne s'agit en aucun cas pour le Gouvernement de « forcer la main » du Parlement ou encore de préjuger de l'adoption du projet de loi sur l'audiovisuel. Il s'agit uniquement de prévoir des dispositions pragmatiques sans lesquelles la Hadopi ne pourra plus fonctionner correctement. Le Gouvernement se félicite donc que ces dispositions aient été maintenues dans le texte de la commission mixte paritaire. Mesdames, messieurs les sénateurs, au moment où s'achève le parcours parlementaire de ces projets de loi, je tiens à vous remercier pour le travail effectué et pour les échanges fructueux que nous avons eus ces dernières semaines.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le 4 février dernier, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur les projets de loi relatifs à l'application de l'article 13 de la Constitution. Ces deux projets de loi, l'un organique, l'autre ordinaire, prévoient, d'une part, d'actualiser la liste des nominations par le Président de la République soumises à l'avis préalable des commissions parlementaires compétentes et, d'autre part, de prolonger le mandat des six membres de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi). Depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V République, le Parlement dispose d'un pouvoir de veto sur certaines nominations effectuées par le Président de la République, « en en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation », comme le prévoit le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Ces nominations sont soumises à l'avis préalable des commissions compétentes de chaque assemblée. Le Président de la République doit y renoncer lorsque l'addition des votes négatifs représente, au total, au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés. Un tel contrôle parlementaire nous paraît indispensable. En effet, l'avis préalable des commissions parlementaires présente un double intérêt. D'une part, il renforce le contrôle des nominations, d'autre part, il garantit la transparence de ces nominations, notamment grâce à l'audition des candidats pressentis. Depuis sa création en 2010, la liste des postes concernés par cette procédure n'a cessé de s'étoffer, constitue une avancée importante en matière de démocratie et de transparence. Les textes adoptés marquent une évolution certaine du champ d'intervention du Parlement. C'est ainsi que, dorénavant, celui-ci se prononcera sur la nomination, par le Président de la République, du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des directeurs généraux de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et, enfin, du président de la Commission d'accès aux documents administratifs. Au total, 55 nominations seront soumises à cette procédure de contrôle. Je me félicite donc des améliorations que les députés et les sénateurs ont apportées à ces deux textes, non seulement des coordinations nécessaires concernant les intitulés des organismes ou des fonctions concernés, mais aussi de l'extension de cette procédure de contrôle à certaines nominations comme

De même, je me réjouis que le rôle de la CADA n'ait pas été minimisé. En effet, cette autorité indépendante joue un rôle fondamental pour garantir les droits des citoyens, moment où la demande d'accès aux documents administratifs n'a jamais été aussi forte. La seule divergence entre nos deux assemblées concernait la SNCF, et plus particulièrement SNCF Réseau. En effet, il aurait été de l'intérêt du Parlement d'intégrer SNCF Réseau dans la procédure prévue par l'article 13, alinéa 5, de la Constitution.

lequel comporte également des dispositions de prolongation des mandats des membres de la En dépit de la technicité apparente de ce qui pourrait être considéré comme une simple série d'ajustements, voire de changements paramétriques, nous touchons en fait à un sujet d'une plus grande importance la fonction constitutionnelle de contrôle du Parlement, telle qu'elle est renforcée depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008. En effet, l'article premier du projet de loi organique modifie la liste des emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du chef de l'État, aux termes de l'article 13 de la Constitution, s'exerce après avis des commissions compétentes de chaque chambre.

Il s'agit donc pour le Parlement d'une garantie, et finalement, d'une sorte de droit de regard. un certain nombre d'organismes sont retirés ou ajoutés à cette liste, tandis que d'autres voient leur nom modifié pour mieux refléter l'évolution de ces structures.

tirent les conséquences d'ordonnances qui n'ont pas encore été ratifiées. Exactement ! On nous dira sans doute que leur ratification éventuelle est une affaire entendue, et qu'il existe un accord plus ou moins large autour de leur contenu, cela ne change rien au fait que, en présentant aujourd'hui ces deux projets de loi, le Gouvernement présume de l'accord futur du Parlement sur d'autres textes. Pour tout dire- vous en conviendrez aisément Nous nous sommes néanmoins prêtés à l'exercice d'autant plus attentivement que le texte aurait initialement fait passer le nombre d'emplois soumis à l'avis préalable des commissions compétentes de 54 à 51. Notre position concernant l'importance du rôle de contrôle du Parlement étant constante, il aurait été incohérent de laisser ce dernier reculer, fût-ce légèrement. Nous avons donc enrichi ces textes en première lecture en incluant dans les emplois soumis à avis le président de la CADA et le directeur général de l'OFII et en sécurisant le rôle de contrôle du Parlement dans ces nominations. La question de l'avis sur le personnel dirigeant des chemins de fer avait en particulier donné lieu à des amendements de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, et ce afin de bien inclure les quatre dirigeants de la SNCF. Nous sommes heureux de constater que les députés ont largement partagé notre vision des choses, en conservant plusieurs de nos apports, et qu'ils ont même ajouté les dirigeants de l'ANSM et de l'Anses à la liste des emplois soumis à la procédure de l'article 13 de la Constitution. Je salue cet heureux mouvement de convergence vers la protection et le renforcement de la fonction de contrôle du Parlement. En revanche, je regrette que nos homologues de l'Assemblée nationale n'aient pas reconsidéré en commission mixte paritaire notre proposition d'inclure le directeur général de SNCF Réseau- ancien établissement public Réseau ferré de France -dans la liste des emplois soumis à l'avis des commissions. La mission particulière de SNCF Réseau en fait, me semble-t-il, un acteur stratégique essentiel au transport en France, et l'y inclure aurait été très judicieux, comme notre collègue Didier Mandelli, rapporteur pour avis, l'avait à l'époque exposé au nom de la commission de l'aménagement du territoire

si le Sénat était opposé à la privatisation de la Française des jeux, la chose étant désormais réalisée, nous avons logiquement fait le choix d'agréer, dès la première lecture, le retrait de son dirigeant de la liste des emplois soumis à la procédure de l'article 13 de la Constitution. En somme, grâce au remarquable travail de nos rapporteurs, ces deux textes finaux me semblent tout

Nous saluons nos collègues députés de La République En Marche, qui n'ont pas suivi la position du Gouvernement, en commission puis en séance, et enfin au cours des travaux de la commission mixte paritaire sur les deux ajouts importants opérés dès le stade de l'examen en commission au Sénat par notre groupe, sous l'impulsion nette de Jean-Yves Leconte, que je salue. Je salue également notre rapporteur pour les avis favorables qu'il a donnés sur deux questions importantes : le président de la Commission d'accès aux documents administratifs et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi été intégrés à la liste des nominations devant relever de cette procédure spéciale. C'est une belle avancée démocratique que nous apprécions tous. Une pierre d'achoppement

filiale de la SNCF. Le rapporteur M. Euzet a fait valoir que « si l'on convenait d'une situation inverse, on établirait une sorte de double légitimité qui pourrait poser des difficultés en termes de gouvernance ». Pourtant, dans la phrase suivante, M. Euzet renvoie sur l'Autorité de régulation des transports pour s'assurer que les décisions de la SNCF respectent l'indépendance de SNCF Réseau. Vous saisissez le paradoxe, paradoxe, sinon la contradiction ! M. Euzet est sans nul doute un juriste reconnu, mais il méconnaît manifestement le nouveau pacte ferroviaire et les intenses discussions qui ont prévalu à ce sujet. J'étais impliqué dans ce débat au cours duquel nous nous sommes collectivement battus, au Sénat, pour transformer huit ordonnances en un véritable texte de loi avec un véritable volet social. Cette question avait pourtant été fort bien expliquée dès la discussion générale du texte par le rapporteur pour avis Didier Mandelli. De trois auditions, nous ne conservons qu'une. Si certains y voient une marque d'intégration du nouveau groupe ferroviaire, nous nous inquiétons de la fragilité de ce que la ministre Élisabeth Borne qualifiait elle-même de « muraille de Chine » qui devait s'ériger entre SNCF Réseau et les autres parties du groupe pour garantir son indépendance à l'heure de la fin du monopole et de l'ouverture à la concurrence. C'est au nom de cette indépendance que nous demandions de garder un droit de regard sur cette nomination, qui aurait permis de mettre de la distance dans la relation hiérarchique évidente entre la SNCF et SNCF Réseau, entre M. Luc Lallemand et M. Cette question de l'indépendance du gestionnaire d'infrastructure est au centre à la fois de nos débats et de l'avenir du système ferroviaire français. Je veux mettre en garde le Gouvernement

Le président de cette autorité, Bernard Roman, a d'ailleurs bien précisé que l'avis préalable des commissions parlementaires serait de nature à accroître l'indépendance et la légitimité des candidats retenus, et plus largement, de l'entreprise SNCF Réseau, en particulier au au regard des autres entités de la SNCF. Permettez-moi de citer mon collègue Jean-Pierre Sueur : « Pourquoi se donner tant de mal pour réduire les pouvoirs du Parlement ? Quel inconvénient y aurait-il à soumettre le directeur général de SNCF Réseau à la procédure du dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution ? Chacun conviendra qu'il n'y avait rien de dramatique à voir chaque groupe politique, au sein des commissions parlementaires concernées, formuler une position. Si le vote devait être négatif, une autre personne serait pressentie. Serait-ce si grave ?

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la commission mixte paritaire est finalement parvenue à un accord, non sans susciter une certaine déception chez ceux qui défendent le maintien d'un réseau de transport de qualité, accessible à l'ensemble des citoyens quelle que soit leur localisation sur le territoire. D'apparence assez anodine, ces textes ont en effet des implications politiques importantes, puisqu'ils définissent les périmètres de contrôle des nominations à des emplois et fonctions clés de notre société pour les libertés, mais également pour le secteur économique. Comme le prévoit le troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution, une grande partie des nominations indispensables à la conduite de la politique du Gouvernement n'est pas soumise au contrôle du Parlement. Cela vaut pour les conseillers d'État, les ambassadeurs, les préfets ou encore les directeurs d'administrations centrales, dont le rôle a pris une importance accrue. Tel n'est pas le cas aux États-Unis, où les ambassadeurs font, par exemple, l'objet d'une audition par le Sénat avant leur prise de fonctions. Le système des dépouilles y est nettement plus étendu, et l'audition parfois d'ailleurs dévoyée à des fins politiques ou politiciennes pour mettre en difficulté le président. L'exercice consiste donc à trouver un équilibre entre la mise en place d'un contrôle parlementaire efficace sur les nominations dans l'intérêt des Français, et la nécessité de garantir des marges de manoeuvre au Gouvernement pour conduire sa politique. Cet objectif justifie que les emplois et les fonctions soumis à ce contrôle parlementaire fassent l'objet d'une liste exhaustive, à condition qu'ils entrent dans l'un des deux cas de figure prévus au cinquième alinéa l'importance pour la garantie des droits et libertés ou pour la vie économique et sociale de la Nation ». Comme l'ont montré nos débats, cette qualification n'est pas toujours consensuelle. Nous avons eu par exemple des échanges animés à propos de la Commission d'accès aux documents administratifs. L'importance de ces fonctions et emplois est susceptible de varier selon l'évolution des compétences attribuées par la loi à ces instances, ou même, plus prosaïquement, en fonction du zèle des personnes nommées. Certaines personnalités ont ainsi marqué durablement leur institution- je pense au Défenseur des droits ou à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. C'est pourquoi il importe d'actualiser régulièrement cette liste, afin qu'elle coïncide pleinement avec l'intérêt général de notre pays- une notion, on le sait, en constante évolution. Dans le champ économique, nos débats ont aussi montré que le contrôle parlementaire est désormais limité par un deuxième obstacle : la remise en cause de l'intervention de l'État dans l'économie. l'économie. Du fait de la privatisation d'entreprises détenues par l'État et de la marginalisation de l'État actionnaire, le pouvoir de nomination étatique disparaît et avec lui, incidemment, le contrôle du Parlement sur ces nominations. relatif à l'importance « pour la vie économique et sociale de la Nation » nous semble encore devoir être précisé : s'agit-il d'une importance systémique, en fonction de la taille, ou alors catégorielle, selon le secteur d'activité ? S'agit-il encore de protéger les monopoles naturels, que certains économistes contestent depuis bien longtemps ? Si l'on comprend facilement qu'il n'est pas utile de maintenir un droit de regard sur les nominations au sein d'entreprises soumises au droit de la concurrence, il paraît néanmoins contestable de priver le Parlement d'un contrôle sur la direction d'entreprises stratégiques pour l'aménagement du territoire, du territoire, dans un contexte où l'égalité et la cohésion des territoires sont devenues des questions prégnantes. C'est justement le cas avec SNCF Réseau. Le groupe du RDSE a toujours abordé la question ferroviaire sans dogmatisme économique, mais, au contraire, avec une forte volonté de pragmatisme et d'efficacité. Peu importent les théories de tel ou tel économiste : notre préoccupation est de lutter contre la dégradation du réseau, notamment celle des petites lignes ferroviaires. Nous pensons donc que si le droit de la concurrence s'oppose à ce que les nominations au sein de SNCF Réseau fassent l'objet d'un contrôle parlementaire, il demeure indispensable de trouver d'autres moyens de renforcer le contrôle du respect par cette entreprise de son obligation de service public sur l'ensemble du territoire de la République. Malgré cette petite dissonance, nous voterons les deux textes. La parole

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi et le projet de loi organique que nous examinons aujourd'hui, tels qu'ils résultent des arbitrages de la commission mixte paritaire, revêtent- je le crois -une double importance pour notre Haute Assemblée.

Les présents textes visent ainsi à modifier et actualiser une loi organique et une loi du 23 juillet 2010 relatives à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution conférant au Parlement un pouvoir de contrôle et d'opposition sur certaines nominations décidées par le Président de la République. Ce contrôle du pouvoir de nomination du chef de l'État, issu de la révision constitutionnelle d'ampleur du 23 juillet 2008 et précisé par le législateur organique en 2010, constitue une avancée pour notre démocratie à plusieurs égards. Tout d'abord, l'audition publique qui précède l'avis de la commission permanente compétente est une garantie de transparence dans l'évaluation des compétences de la personne auditionnée.

dont ces textes ont fait l'objet au cours de la navette illustre bien le travail de coconstruction entre les deux chambres sur un sujet d'une telle importance. Je voudrais aussi saluer l'accord élaboré en commission mixte paritaire, à la construction duquel a contribué notre collègue rapporteur au Sénat Yves Détraigne, que je remercie.

Tout d'abord, les apports importants du Sénat ont été conservés par l'Assemblée nationale et la commission mixte paritaire. C'est le cas de l'extension du champ d'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution à la présidence de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et à la direction générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration C'est également le cas de l'actualisation de l'intitulé de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), ainsi que de l'extension aux membres suppléants de la Hadopi de la prorogation du mandat prévue pour plusieurs membres titulaires. Ensuite, les deux chambres sont parvenues à dépasser leurs désaccords sur la nomination des dirigeants de la SNCF en retenant la rédaction de l'Assemblée nationale. Cette solution n'est pas un échec pour le Sénat. Elle participe au contraire d'une actualisation juridique cohérente en tirant les conséquences, comme le fait le projet de loi organique sur d'autres points, de la transformation de la SNCF en une société unifiée depuis le 1 janvier 2020. commission mixte paritaire de même que le projet de loi organique initial et le texte de l'Assemblée nationale prévoient que seul le directeur général de la SNCF est nommé par le Président de la République après avis du Parlement. Ce dispositif est conforme au droit commun des sociétés détenues directement à plus de 50 % par l'État. Un autre point de divergence résidait dans la nomination à la présidence du conseil d'administration de SNCF Réseau, désormais filiale de la SNCF. La nomination selon la procédure du cinquième alinéa de l'article 13 n'a pas été retenue par la commission mixte paritaire, et ce en cohérence avec le nouveau pacte ferroviaire. Je souhaite, à ce titre, rappeler que le code des transports offre des garanties à l'indispensable indépendance de SNCF Réseau en disposant que « l'Autorité de régulation des transports veille à ce que les décisions de la SNCF respectent l'indépendance de SNCF Réseau ». En tout état de cause, la nomination, le renouvellement et la révocation de ses dirigeants devront faire l'objet d'un avis conforme de l'Autorité de régulation des transports. Enfin, la commission mixte paritaire a utilement prévu la compétence de la commission des affaires sociales pour la nomination de la direction générale de l'Agence Elle a également procédé à une coordination calendaire nécessaire s'agissant de la prorogation des membres de la Hadopi. Finalement, mes chers collègues, les textes de la commission mixte paritaire offrent un équilibre pertinent. En portant à 55 le nombre de postes soumis à la procédure de nomination du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, il confirme et conforte le pouvoir de contrôle du Parlement, tout en garantissant la cohérence de notre ordonnancement juridique. Pour toutes ces raisons, et en saluant de nouveau le travail de conciliation accompli, notamment par M. le rapporteur, le groupe La République En Marche votera ces deux textes.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le 17 décembre dernier, par ma voix, le groupe CRCE a exposé les raisons de son opposition à ces projets de loi organique et ordinaire. Nous avions rappelé alors alors les limites du contrôle parlementaire des nominations proposées par le Président de la République. En effet, la nécessité de recueillir trois cinquièmes de votes contre au sein des deux commissions concernées, à l'Assemblée nationale et au Sénat, limite considérablement ce pouvoir de contrôle. Nous avons toujours proposé l'inverse : exiger trois cinquièmes de votes positifs supposerait un vrai consensus sur ces nominations. À l'occasion des débats dans les deux chambres, y compris en commission mixte paritaire, beaucoup se sont émus d'une certaine violence faite au Parlement, ce qui est malheureusement monnaie courante ces temps-ci, avec la référence à des ordonnances concernant la nouvelle organisation de la direction de la SNCF. En effet, le Parlement est censé élargir son contrôle sur des nominations concernant des postes dont la création par ordonnance n'a même pas été ratifiée, Comment ne pas penser, dans ces conditions, au projet de loi sur les retraites, qui comprend vingt-neuf habilitations à légiférer par ordonnance ? Le Gouvernement dit au Parlement : « Ne vous inquiétez pas, vous les ratifierez.

C'était le cas en 1945 ou en 1958. Aujourd'hui, selon nous, rien ne justifie démocratiquement le recours à un tel autoritarisme constitutionnel. parce qu'il est temps de faire respecter les droits des assemblées, nous pensons qu'il faut vite rééquilibrer les pouvoirs entre exécutif et législatif. Or ce n'est certainement pas en acceptant de perpétuer la soumission au pouvoir présidentiel de nomination, cadre dans lequel ce texte s'inscrit, s'inscrit, que nous irons dans le sens de la réhabilitation des pouvoirs parlementaires. Nous faisons donc entendre une voix dissonante dans cet hémicycle ce soir en confirmant notre vote contre ces deux textes, même si je tiens à saluer le travail du rapporteur et de nos collègues de la commission des lois. La parole

C'est grâce à elle que nous sommes amenés à examiner une liste de nominations, qui sont donc soumises à l'avis préalable de nos commissions.

pour la transparence de la vie publique. C'est aussi un contrôle qui est effectué de manière bienveillante. Nous savons tous qu'il n'y a jamais eu d'opposition manifestée à l'égard d'une nomination proposée par le Président de la République.

en cas de cohabitation, avec, par conséquent, des répartitions de majorité différentes, même si, encore une fois, pour ne pas retenir une proposition du Président de la République, la majorité à réunir est assez forte.

Nous connaissons la solution qui a été retenue, seul le directeur général de la SNCF restant soumis à ce contrôle. Cela ne me choque pas pour une autre raison, qui n'est plus juridique, mais qui est tout simplement lié

à une réduction du nombre des autorités administratives indépendantes, pas forcément par disparition, mais au moins par fusion. Nous sommes toujours étonnés par un phénomène extraordinaire que nous observons dans nos propres conseils municipaux quand un élu municipal siège dans un syndicat : par une mutation tout à fait étonnante,

nous ne cesserons pas de dire qu'il faudrait réduire le nombre de ces autorités, tout en appréciant que le contrôle parlementaire sur les nominations puisse être un jour renforcé. En résumé, pour le groupe centriste, il faut moins d'autorités administratives indépendantes et plus de désignations La discussion générale commune est close. Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale les textes élaborés par les commissions mixtes paritaires, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble